Initiés par le Président Chirac en 2003, ces sommets permettent de renforcer le rôle de la France et la place de ses collectivités du Pacifique dans cette région océanienne que le Président Emmanuel Macron englobe désormais dans l'axe indopacifique, comme il l'a évoqué dans ses discours à Sydney et à Nouméa en mai 2018. Cet élargissement stratégique entraînera-t-il un nouveau format du sommet ? Pour l'heure, nous ne savons presque rien sur le cinquième sommet. Aura-t-il bien lieu cette année ? À quelle date ? Le Président de la République s'y rendra-t-il ? Sa présence est symboliquement indispensable. Le quatrième sommet a eu lieu à Paris juste avant la COP21 ; le climat en fut le thème principal. Les chefs d'État et de gouvernement présents, conscients que leur région est celle où le plus grand nombre d'États pourraient disparaître à cause du réchauffement, se sont battus pour la limitation à 1,5 degré au lieu de 2 Le cinquième sommet France-Océanie interviendra à l'approche d'échéances majeures en matière de biodiversité. Ne pourrait-il alors être l'occasion non seulement de faire un bilan des objectifs de la COP21, mais aussi de mobiliser la communauté internationale sur la biodiversité, notamment sur la question des aires marines protégées, qui est au coeur des préoccupations des États du Pacifique Notre pays a un rôle à jouer en Océanie où s'exprime un désir de France certain et où il sera, après le Brexit, le seul pays européen présent. Il y contribuera à la promotion des valeurs démocratiques, au maintien de la paix et à la lutte contre les tentations hégémoniques. Le cinquième sommet sera-t-il le lieu et le temps le lieu et le temps d'une explication plus complète de la stratégie de l'axe indopacifique ? La parole

a déjà participé en mai dernier à un dialogue de haut niveau avec un certain nombre de chefs d'État et de gouvernement des États insulaires voisins des territoires ultramarins concernés, et il a souhaité pouvoir tenir un cinquième sommet France-Océanie.

Les Républicains. Ma question s'adresse à Mme la ministre des solidarités et de la santé. Madame la ministre, lundi matin, la France, la région Occitanie, le département de la Haute-Garonne et particulièrement la ville du Lherm se sont réveillés sous le choc. Je souhaite d'abord apporter tout mon soutien et ma compassion aux familles endeuillées. Ce que redoutaient toutes les personnes concernées par la dépendance et par l'accueil réservé à nos aînés venait de se produire

Je ne reviendrai pas, madame la ministre, sur la chaîne de dysfonctionnements qui a conduit à ce désastre humain. Laissons la justice faire son travail. Vous avez insisté sur votre volonté de comprendre les causes de ce drame et de tirer les enseignements de ces tragiques événements.

le manque cruel d'effectifs, sur l'absence de revalorisation des métiers du grand âge et des rémunérations, et sur l'épuisement du personnel, qui, régulièrement, en se mettant en grève, tente d'alerter sur les rythmes de travail et dénonce les conditions de prise en charge de nos aînés. L'humain n'est plus au coeur de notre mission d'accompagnement des personnes âgées, alors même que certains Ehpad génèrent des profits substantiels. Madame la ministre, ma double question est simple. Le rapport Libault sur le grand âge et l'autonomie, qui vient de vous être remis, avance un certain Quand seront-elles mises en oeuvre ? Quels seront les financements dédiés ? L'urgence est là, nous ne pouvons plus attendre

sensibles au drame survenu dans la nuit de dimanche à lundi dans un Ehpad de votre département. Je m'y suis rendue mardi pour rencontrer les familles des victimes et les personnes qui ont été hospitalisées, ainsi que le personnel, également très choqué. D'après les

Contrairement à ce que beaucoup de personnes pensent, les forêts ne sont pas immuables. Elles sont vulnérables et requièrent toute notre attention. Les forêts dont nous profitons à ce jour sont le fruit des choix et du travail des générations passées.

Face à ces usages multiples de la forêt et du bois, face aux changements climatiques, vous le savez, monsieur le ministre, la forêt a besoin en urgence d'une politique forestière volontaire et d'un fonds stratégique alimenté à la hauteur des besoins. Fragilisées depuis plusieurs mois par des déficits hydriques et des températures particulièrement clémentes, nos forêts sont victimes d'attaques de parasites et subissent des crises sanitaires d'ampleur. Le sujet pourrait paraître secondaire, sauf qu'il concerne déjà plus de 1 million de mètres cubes d'essences résineuses, soit 30 % de la récolte annuelle dans les seules régions Bourgogne-Franche-Comté et Grand Est. Toute l'Europe du Nord est touchée, ce qui risque d'engorger les marchés, de faire chuter les cours, de mettre en difficulté nos entreprises et de déstabiliser durablement l'approvisionnement de secteurs stratégiques ; je pense à la construction, secteur pour lequel la France importe déjà. Au-delà des pertes économiques, estimées à 71 millions d'euros en Bourgogne-Franche-Comté et dans le Grand Est, l'impact environnemental lié aux risques d'incendie ou aux coupes rases sur des milliers d'hectares est également majeur. Monsieur le ministre, pour enrayer ces phénomènes, les professionnels de la filière attendent en urgence de votre part la mise en place d'un plan de transport longue distance permettant d'évacuer rapidement les bois scolytés des régions productives vers les régions demandeuses, et ce avant

De façon plus générale, j'ai conscience que cette menace inédite crée une inquiétude dans toute la filière. L'intensité des dommages occasionnés par les scolytes sera largement tributaire des conditions météorologiques de ce printemps. Pour calibrer au mieux la réponse que nous devons apporter à cette crise, il faut d'abord disposer d'un état des lieux précis. C'est pourquoi le ministère de l'agriculture et de l'alimentation a organisé et financé, depuis l'automne dernier, un état des lieux complet par télédétection sur les deux régions que vous avez évoquées. Les premiers résultats de cette enquête ont été portés à la connaissance de l'ensemble des acteurs de la gestion et de l'exploitation forestière des régions concernées. Le but est de leur permettre de mieux cibler leur action et d'accélérer la dynamique de récolte des bois attaqués afin d'enrayer la propagation des scolytes. Ces premiers résultats permettent de localiser les peuplements qui étaient attaqués à l'automne. Une prochaine mise à jour de cette cartographie permettra d'apprécier les évolutions de l'atteinte des peuplements d'épicéa au début du printemps. Au-delà de ces mesures d'observation, les services de nos ministères étudient actuellement le cadre dans lequel pourraient être mises en place des mesures

Aujourd'hui, en France, on estime qu'environ 700 000 personnes vivent avec le spectre de l'autisme, dont 100 000 enfants. Il n'y a qu'assez peu de temps que ce trouble est correctement diagnostiqué. Par conséquent, les patients étaient souvent mal accompagnés jusqu'alors. Nous avons tous dans notre entourage des parents d'enfants, d'adolescents ou de jeunes adultes démunis face à la difficulté de vie ou de communication de leur enfant. J'ai en tête l'exemple d'une jeune femme, Éva, dont le diagnostic Asperger, une des diverses formes de l'autisme, ce syndrome prenant lui-même des formes multiples, a été posé très tardivement. Jusqu'à ce diagnostic, elle qualifiait ses relations sociales d'enfer. Je reprends ses mots : « L'autisme seul a ses bons côtés et ses mauvais, et je ne le vois pas du tout comme un handicap, mais plutôt comme une différence. C'est avec les autres que ça devient un handicap, un enfer. Pourtant, il a fallu commencer par ce diagnostic et ce constat, et donc par sa prise en charge pour que la vie de cette jeune femme change. Après un parcours scolaire et professionnel chaotique-vendeuse dans un commerce de bouche avec une relation clientèle difficile-, difficile-, elle a été reçue fin 2018 à Grenoble École de Management pour suivre la formation Data Asperger. Elle se dit enfin « soulagée et heureuse d'être considérée en tenant compte de ce syndrome Nous serons amenés à discuter prochainement de l'inclusion des enfants en situation de handicap dans le projet de loi pour une école de la confiance. Il sera essentiel de réfléchir à la prise en compte spécifique des élèves autistes. Il me semble aujourd'hui nécessaire, un an après le lancement de la stratégie nationale pour l'autisme pour les années 2018 à 2022, de nous faire part des avancées de ce plan, évidemment pour les aspects relatifs à la scolarisation de ces enfants, mais aussi pour le diagnostic et l'intervention précoces. De nombreuses personnes sont, hélas ! concernées. Il faut conclure ! Pouvez-vous, madame la secrétaire d'État, nous éclairer sur ce sujet ?

Buis, un point d'étape est important, car nous avons souscrit le 6 avril de l'année dernière à cinq engagements dans le cadre de la stratégie nationale pour l'autisme au sein des troubles du neuro-développement, pour une enveloppe de 344 millions d'euros nouveaux. Ces engagements sont portés par une conviction, celle de mobiliser la recherche et la science. Notre objectif est de faciliter le parcours de vie des personnes avec autisme et de leur famille. Il s'agit surtout d'un engagement de responsabilité collective du Gouvernement. Nous nous engageons d'abord sur une action résolue en faveur du repérage et du diagnostic précoce des troubles neuro-développementaux, parmi lesquels l'autisme. Avec Agnès Buzyn, nous investirons massivement 90 millions d'euros d'ici à 2022 pour prévenir, dès les premiers âges, les sur-handicaps

au milieu des autres. Enfin, nous améliorons la pertinence des accompagnements des personnes adultes en les diagnostiquant, ainsi qu'en prévoyant un parcours inclusif vers le logement et l'emploi.

le Président de la République avait indiqué qu'il fallait « renforcer la déconcentration pour adapter les politiques de l'État aux territoires ». Le 21 mars, M. le ministre Darmanin a déclaré, pour sa part, vouloir « mobiliser davantage de fonctionnaires au plus près du terrain Je ne vous cache pas, monsieur le ministre, que cette perspective, en théorie, nous va droit au coeur tant il nous paraît indispensable que les services publics d'État puissent être pleinement déployés et tant il nous paraît indispensable également que ces fonctionnaires puissent être mieux identifiés afin de les mobiliser facilement chaque fois que c'est nécessaire. la dématérialisation n'est pas la seule réponse possible. Il est temps aujourd'hui que nos concitoyens comme leurs représentants, les élus, puissent apprécier la réalité de cette déconcentration, pleinement partenaire d'initiatives locales démultipliées. Or, en tant qu'élus de la République, que constatons-nous ? Nous constatons que des fonds ne sont pas consommés ou sont souvent mobilisés par les mêmes, faute d'une ingénierie suffisante pour décrypter les circulaires. Notre collègue Maryse Carrère avait ainsi pointé du doigt sur nos travées la sous-consommation dramatique de fonds européens et leur possible annulation à hauteur de centaines de millions d'euros. Nous constatons que des collectivités locales, faute d'interlocuteurs d'État, font appel à des cabinets privés afin d'éviter des contentieux lourds. Nous notons que les préfectures et les sous-préfectures n'accompagnent plus assez, comme elles le devraient, les maires et communautés de communes tout au long des procédures d'application des normes, et pire encore dans la quête tortueuse des demandes de subventions ! Mes chers collègues, vous ne me démentirez pas, combien d'élus nous disent qu'ils ont besoin d'être accompagnés en amont de manière directe et concrète, réactive et proche des réalités ! Monsieur le ministre, il est temps de redonner du lustre à la présence territoriale de l'État comment comptez-vous mieux mobiliser le maillage territorial de l'État et redonner ainsi du souffle aux initiatives locales, et ce dans tous les territoires et pour toutes les communes ? La parole

pour renforcer les infrastructures, mais aussi les usages du numérique. Le deuxième point que vous soulignez et auquel je suis profondément attaché concerne le volet accompagnement. L'État doit être un acteur qui accompagne les collectivités. C'est fondamentalement

Les nombreuses actions organisées aujourd'hui-il y en a en ce moment même-en témoignent. La création des établissements publics des savoirs fondamentaux cristallise les mécontents. Concevoir un établissement unique école-collège, sous gouvernance de ce dernier, c'est porter une attaque sans précédent à l'école. Très bien ! Dans ces établissements, les directeurs d'école disparaîtraient au profit de chefs d'établissement et d'adjoints davantage missionnés pour gérer la pénurie de moyens que pour porter un projet pédagogique et accompagner les élèves. Peu de chance qu'ils aient le temps d'échanger avec les parents à la grille de l'école ou d'assumer les tâches multiples qui contribuent à la réussite des enfants dans des établissements XXL ou multi-sites. Mais surtout, au prétexte d'un vague intérêt pédagogique, on pourrait rationaliser, mutualiser, regrouper les écoles avec des conséquences graves : de gros établissements éloignés des familles portant le coup de grâce aux écoles rurales. Les fermetures de classes, injustifiées, qui se multiplient dans nos territoires et conduisent à des effectifs surchargés ne suffisent-elles donc plus ? Vous faut-il passer à la vitesse supérieure Ce n'est pas ce que veulent nos concitoyens ! Faut-il que vous soyez sourd pour ne pas entendre la demande de proximité qui s'exprime comme jamais dans le pays, grand débat ou pas ? Monsieur le ministre, ma question est donc simple : renoncerez-vous à la création de ces établissements publics des savoirs fondamentaux,

Monsieur le ministre, vous venez de lancer un appel à la mobilisation, je pense qu'il sera entendu ! Elle a raison ! Nous avons l'expérience sur le terrain

de la santé. Mardi dernier, le 2 avril, un hommage était rendu à Paris aux morts de la rue. Chez nous, en France, en 2018, 566 sans-domicile sont morts dans la rue.

Ils sont morts, trop souvent dans l'indifférence, sur la voie publique, dans des abris de fortune-parking, cage d'escalier, cabane de chantier ...-, parfois dans un lieu de soins ou une structure d'hébergement. Ils ne font que trop rarement la une de l'actualité, mais c'est la cruelle réalité d'aujourd'hui, dans notre France, pays des droits de l'homme ou, comme Robert Badinter le précisait, « plutôt la France de la Déclaration des droits de l'homme La responsabilité est collective. Elle perdure depuis déjà de trop longues années. Et ce qu'il y a de scandaleux dans le scandale, c'est qu'on s'y habitue. Madame la ministre, un véritable plan d'extrême urgence s'avère indispensable pour ne pas avoir à constater, dans un an, la triste réalité des chiffres de 2018. Permettez-moi, mes chers collègues, de m'adresser à nous tous également. Notre Haute Assemblée peut aussi avoir la noble ambition d'être le porte-voix de ces sans-voix. C'est une ambition à porter, un défi à relever. À ce moment de mon propos, je veux remercier le travail remarquable de l'ensemble des associations caritatives et humanitaires pour leur attention scrupuleuse et leur indispensable action. Sans elles, notre pays connaîtrait un véritable raz-de-marée de la misère. Notre illustre prédécesseur Victor Hugo écrivait : « L'homme est fait non pas pour traîner des chaînes, mais pour ouvrir des ailes. » Brisons, mes chers collègues, les chaînes de l'indifférence et écoutons respectueusement le silence de ces 566 sans-abris qui nous ont quittés l'an passé. La parole

Il faut continuer avec énormément de détermination. Victor Hugo écrivait aussi, dans une de ses correspondances : « Pour moi, l'idée de nation se dissout dans l'idée d'humanité. » La grandeur d'une nation se mesure à cette humanité, à cette solidarité qu'elle est capable d'octroyer aux plus fragiles. Soyez assuré, monsieur le sénateur, que nous continuerons d'agir non seulement avec beaucoup de force et d'humilité, mais surtout avec détermination face au sans-abrisme.

d'ici à la fin du quinquennat, plus personne ne paiera la taxe d'habitation, sans augmentation d'impôt, a martelé le Président de la République. Depuis cette annonce, non concertée, les élus attendent vos propositions, le dégrèvement étant, pour l'heure, financé par du déficit et, donc, par de la dette. En octobre dernier, on « balançait » son maire avec mépris. Quelques semaines plus tard, les élus de proximité étaient devenus le rempart de notre démocratie, un pilier sur lequel le Gouvernement souhaitait s'appuyer. Alors que les communes votent aujourd'hui leur budget, et à moins d'un an des municipales, les élus ont besoin de lisibilité, de stabilité et de confiance sur l'évolution de leurs ressources pour programmer leurs projets.

obérant quelque peu vos projections financières-nous savons ce qu'il advint de la fiscalité écologique qui devait venir au secours du financement du dégrèvement ... Le ministre de l'action et des comptes publics a indiqué à l'Assemblée nationale que la suppression de la taxe habitation pour tous était confirmée, hors résidences secondaires. des logements vacants et des bases locatives

Ma question est simple : comment envisagez-vous de financer votre réforme, dans le respect de la libre administration des collectivités, aucune de vos hypothèses n'ayant jusqu'alors tenu la corde ? Pour conclure, monsieur le Premier ministre, je ferai miens les propos de notre président, Gérard Larcher : « On ne redressera pas notre pays sans les élus et les territoires. » Ne l'oubliez pas

supprimer la taxe d'habitation pour l'ensemble des résidences principales, et non pour les résidences secondaires, comme nous l'avons dit depuis le début. Nous veillerons à ce que l'intégralité des recettes perçues par les collectivités, communes et intercommunalités soit compensée.

d'une réforme importante, monsieur le sénateur, dont les enjeux sont majeurs. Nous travaillerons à la compensation des recettes pour les collectivités, sans créer d'impôts nouveaux,

En 2018, j'alertais par courrier M le ministre de l'intérieur sur la non-application du critère des centres d'intérêt matériels et moraux, dits CIMM, dans les règles de mutation de la police nationale. Le 5 février dernier, je recevais une réponse m'indiquant qu'il avait été « demandé au préfet, directeur général de la police nationale, de faire procéder à un examen attentif de ma demande Le Conseil d'État a été, semble-t-il, plus prompt que les services de l'intérieur en apportant une réponse définitive à ma question. Dans un arrêt du 18 mars dernier, il donne raison à un fonctionnaire du corps de la police nationale qui contestait la circulaire du ministre de l'intérieur sur les mouvements de mutation des agents du corps d'encadrement et d'application de la police nationale. Cet arrêt est sans ambiguïté : dès l'application de la loi, l'administration doit tenir compte des CIMM dans l'examen des demandes de mutation. Monsieur le secrétaire d'État, cet arrêt du Conseil d'État s'applique à l'ensemble de la fonction publique, dans l'ensemble des territoires ultramarins, où la non-prise en compte des CIMM est quasi généralisée. généralisée. Nous, parlementaires, députés et sénateurs, sommes régulièrement sollicités par des fonctionnaires ultramarins considérant que leur demande d'affectation dans leur territoire d'origine a été injustement refusée, qu'il s'agisse de la police nationale, de l'administration pénitentiaire ou de l'éducation nationale. Aussi, je vous demande si les décisions d'affectation des fonctionnaires ultramarins pour l'année 2019 vont bien être revues par l'ensemble des administrations en prenant en compte l'arrêt du Conseil d'État du 18 mars dernier. La parole

dont bénéficient les fonctionnaires d'origine ultramarine dès lors qu'ils peuvent justifier de ce centre d'intérêt matériel et moral en outre-mer. Il s'agit d'une notion récente : jusqu'en 2017, son application était extrêmement disparate, voire inexistante dans un certain nombre de corps.

nombre de situations. À ce stade, 11 % du volume total des demandes de mutation était accompagné de la demande de reconnaissance d'un centre d'intérêt matériel et moral. 25 % des mutations vers les territoires d'outre-mer ont été effectuées en application de cette priorité légale d'affectation, liée à la justification d'un CIMM. Enfin, 75 % des demandes de mutation vers les outre-mer

des mutations qui permettent le retour vers les territoires ultramarins, nous travaillons aussi à la mise en place de concours nationaux à affectation locale, de manière à rendre possible l'adaptation des politiques de recrutement aux besoins des territoires. Prochainement, un décret sera soumis à la concertation, avant de passer en Conseil d'État.

Le week-end dernier, non loin de Toulouse, une vingtaine de résidents de l'Ehpad La Chêneraie auraient été victimes d'une grave intoxication alimentaire : 17 d'entre eux ont été hospitalisés, et 5 ont perdu la vie. Au-delà de la colère légitime des familles et des proches, nous ne pouvons rester insensibles à ce drame, comme s'il s'agissait d'un simple fait divers. Madame la ministre, vous êtes à la tête d'un grand ministère, avec d'énormes responsabilités, et vous avez notamment la charge de protéger les publics vulnérables. Nous ne mettons nullement en cause votre implication au quotidien pour remplir au mieux vos missions : vous le faites avec conviction, confiance et rigueur. Mais un tel drame interroge forcément l'opinion publique et les parlementaires, car nous sommes nombreux à compter un ou plusieurs Ehpad dans nos territoires. Avec toutes les réserves d'usage, une enquête étant en cours, pouvez-vous nous éclairer sur l'état d'avancement des investigations ? D'après les dernières informations parues dans la presse aujourd'hui, les personnes seraient pour la plupart décédées par étouffement consécutif aux vomissements. Par ailleurs, quelles actions le Gouvernement envisage-t-il pour rassurer les parents et les pensionnaires en Ehpad afin de garantir une meilleure sécurité et une meilleure surveillance de ces résidents ? La

alimentaire. Je tiens à rappeler l'engagement du Gouvernement sur un grand plan dédié à la prise en charge des personnes âgées et de la dépendance, que nous proposons de traduire par une loi d'ici à la fin de l'année.

Piveteau souligne la nécessité de mieux former les professionnels et de leur donner des outils pour être bien-traitants auprès des plus vulnérables. Nous sommes totalement engagés pour travailler à une feuille de route

remercie de toutes ces précisions, madame la ministre. S'il est vrai que le risque zéro n'existe pas, nous devons tout faire pour éviter de tels drames et, surtout, tout mettre en oeuvre pour que les pensionnaires des Ehpad soient encore mieux accompagnés et encadrés.

la France réalise des efforts importants pour assurer une formation d'excellence à nos futurs médecins et ainsi garantir la qualité des soins dispensés à nos compatriotes. Ce sont les établissements d'enseignement supérieur publics qui réalisent logiquement cette formation. Elle est donc légitimement gratuite. Le coût moyen de formation d'un étudiant est estimé à environ 150 000 euros sur toute la durée de son cursus. L'État et les collectivités investissent ensuite massivement pour inciter les médecins à s'installer dans les territoires qui en ont le plus besoin. L'an passé, je vous avais demandé un état des lieux de l'ensemble de ces dispositions et de leurs coûts pour la puissance publique, sans jamais avoir obtenu de réponse. Madame la ministre, comment expliquer à nos concitoyens et aux élus locaux avec autant d'investissement, à doter les territoires ruraux, mais aussi périurbains sensibles, de médecins en nombre suffisant ? À Morlaix, à une heure du CHU de Brest, comment comprendre que le service de cardiologie de l'hôpital public ait fermé ses portes, faute de cardiologue, alors que la clinique privée de la ville a opportunément développé son offre de consultations cardiologiques ? Comment expliquer qu'on laisse s'installer des médecins dans des zones déjà sur-dotées sans utiliser le levier du déconventionnement ? Comment expliquer que, malgré toutes les mesures incitatives, nous n'arrivions pas à les faire s'installer là où il y a un réel besoin ? Madame la ministre, ma question est simple : allez-vous rendre public le coût de l'ensemble des dispositifs d'aides à l'installation des médecins ? Allez-vous décider de déconventionner les médecins qui s'installeraient en zones denses et prendre des mesures coercitives à leur encontre pour qu'ils s'installent dans les zones sous-dotées ? La parole

de s'engager dans les territoires en favorisant l'exercice pluriprofessionnel et les délégations de tâches avec d'autres professionnels de santé-notamment autour des pathologies chroniques-, en leur permettant de récupérer du temps médical grâce à des assistants médicaux. Il s'agit des consultations avancées de spécialistes qui viennent des hôpitaux publics, ou même du secteur libéral, et de développer ces consultations itinérantes sur le territoire. Nous souhaitons également redonner de la place dans les hôpitaux de proximité aux médecins généralistes qui visent des exercices diversifiés. C'est une politique incitative, mais pas uniquement financière, loin de là. Nous voulons pérenniser dans les territoires les médecins qui ont envie d'y être et qui prennent du plaisir à soigner les malades. C'est la politique que je mène. Nous sommes beaucoup interpellés sur la coercition et sur les mesures qui pourraient obliger les médecins à s'installer. Malheureusement, comme vous le savez, nous souffrons d'une démographique médicale catastrophique, qui n'a pas été anticipée. Nous avons quelques années difficiles devant nous. Aujourd'hui, il n'y a plus de zones sur-denses en France. Il n'y a plus de zones

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, les missions locales font partie intégrante du service public de l'emploi pour les jeunes de 16 à 25 ans.

logiques de bassin, fusions, baisse des subventions de fonctionnement, financement des appels à projets, mise en place d'un bonus-malus, et cela sans concertation avec le réseau des missions locales, acteurs indispensables dans les territoires pour l'emploi de nos jeunes. En dépit de la diversité des personnes accueillies, dont certaines sont déjà exclues de tout autre dispositif ou structure, ce sont plus de 1 million de situations professionnelles qui ont été mobilisées pour les jeunes par les missions locales, dont 544 000 contrats de travail-en de 3 % sur un an-, 40 000 contrats en alternance-en augmentation de 8 % sur un an-et 16 000 retours en formation-en hausse de 7 %. Les missions locales doivent leur réussite à un accompagnement global et personnalisé du public concerné et à une expertise de leur territoire et de son contexte économique. Mais n'oublions pas que les missions locales ce sont également des équipes, dont l'inquiétude s'accroît en raison d'une absence de lisibilité de leur devenir. Monsieur le ministre, ce manque de confiance dans leur avenir crée une tension sociale dans le réseau. Quelles sont

rester dans son rôle. Le ministère du travail participe au budget des missions locales à hauteur de la moitié, le reste étant financé par les collectivités-agglomérations, communautés de communes, départements ou régions. Nous souhaitons aller vers une approche de résultat. Aujourd'hui, nous subventionnons le fonctionnement et l'activité liés à la garantie jeunes. Or la notion de résultat n'est pas liée à la dépense de fonctionnement. Nous voulons donc qu'une partie de la subvention soit liée au résultat.

encouragement au résultat, voilà le sens que nous voulons donner à la politique et le sens et la place que nous voulons donner aux missions locales !

Monsieur le ministre, depuis 140 ans, Belfort forge une des plus belles aventures industrielles de notre pays : il s'agit notamment des centrales nucléaires et du TGV. Ce savoir-faire est aujourd'hui gravement menacé par la situation du site de General Electric à Belfort. Lors du rachat de la branche énergie d'Alstom, le projet de GE, soutenu par le Gouvernement, prévoyait la création de 1 000 emplois nets en France. Le ministre de l'économie et des finances de l'époque, l'actuel Président de la République, était d'ailleurs venu à Belfort. Permettez-moi Belfort a un avenir industriel. Cet avenir industriel fait partie d'abord des engagements pris de part et d'autre, et ces engagements sont suivis par le Gouvernement. » Depuis, nous avons assisté à la suppression de 264 postes et à la non-création des 1 000 emplois promis. gaz, près de 1 000 postes seraient aujourd'hui menacés. L'annonce de ce plan social aurait été opportunément repoussée pour ne pas intervenir avant les élections européennes. Si tel est le cas, l'économie du Territoire de Belfort et les salariés de GE méritent mieux que des arrangements politiques. Seul le Gouvernement dispose des clés pour amorcer le redressement de l'industrie belfortaine.

C'est aussi le marché très porteur des moteurs d'avions porté par Safran et General Electric Aviation. C'est encore l'implantation de l'Institut national de stockage d'hydrogène ou l'appel à projets « Territoires d'innovation

Le 7 février dernier, Bruno Le Maire et moi-même réunissions le comité de suivi des engagements pris par GE lors de l'acquisition de la branche énergie d'Alstom. Nous avions alors pu constater les engagements et les actions pris par GE-Alstom. Entre 2015 et 2018, l'investissement s'est élevé à près d'un milliard d'euros

des énergies fossiles. Elle est actuellement en train de revoir son modèle économique dans le monde entier. Dans ces conditions, nous ne restons pas les bras ballants. Nous avons mis en place un fonds de réindustrialisation, abondé par GE à hauteur de 50 millions d'euros, qui sera présidé par un expert industriel, associera les élus et examinera les projets industriels que vous avez mentionnés. En effet, il ne suffit pas d'avoir de bonnes idées, encore faut-il les mettre en oeuvre de manière professionnelle. Par ailleurs, nous sommes ailleurs, nous sommes attentifs à la réorganisation de GE, et nous saluons positivement le renforcement de GE Renouvelable, qui représente 40 000 employés dans le monde

Nous accompagnerons donc GE, mais dans un avenir qui ne sera pas fondé sur les énergies fossiles. Nous en

de la proposition de loi tendant à sécuriser l'actionnariat des sociétés publiques locales et des sociétés d'économie mixte, présentée par M.

La séance est reprise. Mes chers collègues, par lettre en date de ce jour, le Gouvernement a demandé le retrait de l'ordre du jour du mardi 9 avril de l'examen en nouvelle lecture de la proposition de loi portant création d'une Agence nationale de la cohésion des territoires et de la lecture des conclusions de la commission mixte paritaire sur la proposition de loi organique relative à la nomination du directeur général de l'Agence nationale de la cohésion des territoires. Il a également demandé le retrait de l'ordre du jour du mercredi 10 avril de la suite de l'examen en nouvelle lecture du projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises.

mes chers collègues, les établissements publics locaux jouent un rôle particulièrement actif dans l'économie locale. Actuellement, on en dénombre environ 1 300, employant au total 70 000 salariés. Ils génèrent un chiffre d'affaires de près de 14 milliards d'euros. Grâce à l'évolution législative, les collectivités locales ont pu s'adapter aux exigences liées aux enjeux en matière d'aménagement, d'équipements et de logements. Il existe ainsi une ingénierie publique qui offre aux élus locaux une palette de dispositifs conjuguant la nécessité du cadre administratif et la performance économique. Grâce à l'expérience de nos parcours d'élus locaux, nous savons tous combien les sociétés d'économie mixte, les SEM, les SEM à opération unique, les SEMOP, ou encore les sociétés publiques locales, les SPL, sont particulièrement utiles pour mener à bien des opérations qu'une seule collectivité ne serait pas en mesure de mener. Cette souplesse juridique a en outre le mérite d'accélérer la prise de décision. Mutualisation, coopération, innovation et maîtrise des budgets font partie intégrante du « logiciel » des élus locaux, qui ont trouvé de nouvelles formes de coopération et de gouvernance grâce aux dispositifs de l'économie mixte. Car, ce qui nous anime, c'est bien la mise en oeuvre de projets pour les territoires et pour leurs habitants ! Plus généralement, les EPL, les entreprises publiques locales, peuvent être considérées comme une « boîte à outils » facilitant la mise en oeuvre des politiques publiques locales, notamment en matière d'urbanisme. La société publique locale issue de la loi Raoul du 28 mai 2010 est venue compléter cette palette. La SPL s'impose dès lors comme un outil de coproduction entre plusieurs niveaux-communal et intercommunal- et organise la maîtrise d'ouvrage publique. Cette loi a permis de renforcer la capacité d'action des collectivités. Je rappelle que, à cette époque, la France était encore le seul pays de l'Union européenne où il n'était pas encore possible pour les élus locaux de créer de telles entreprises. Le code général des collectivités territoriales s'est donc enrichi voilà environ neuf ans de l'article L. 1531-1, qui dispose que les communautés et leurs communes peuvent constituer une SPL uniquement « dans le cadre des compétences qui leur sont attribuées par la loi Ainsi une collectivité territoriale ne pourra-t-elle pas faire faire par une SPL ce qu'elle ne pourrait pas faire elle-même. Pour autant, un arrêt du Conseil d'État du 14 novembre 2018 a suscité des inquiétudes légitimes dans le secteur de l'économie locale et des collectivités. En effet, le Conseil d'État a eu une interprétation particulièrement restrictive du lien de compatibilité entre, d'une part, les compétences des collectivités ou de leurs groupements actionnaires d'une SPL et, d'autre part, l'objet social de cette SPL. En résumé, cet arrêt remet en cause la possibilité pour des collectivités de niveaux différents d'être actionnaires de la même SPL. Pourtant, c'est bien cette dimension qui fait toute la pertinence d'une

Il est uniquement question dans ce texte de lever une incertitude juridique et de sécuriser la possibilité, pour des collectivités locales de strates différentes, d'être actionnaires de la même EPL. Ni plus ni moins En effet, le texte de la loi étant insuffisamment précis et certains arrêts rendus contradictoires, il convenait de clarifier l'intention du législateur. Il était urgent de réagir, car bon nombre de maires et dirigeants d'EPL ont déjà reçu des préfectures une circulaire les incitant à mettre en conformité leur actionnariat dans les meilleurs délais, soit avant le 8 décembre 2019. Ainsi 200 à 300 structures seraient-elles dans le viseur. Il serait désagréable que la ville de Vernon, le département de l'Eure et Seine Normandie Agglomération ne puissent plus être actionnaires ensemble de la SPL Campus de l'Espace.

et la communauté d'agglomération Pau Béarn Pyrénées ne puissent plus être actionnaires ensemble des SPL Palais Beaumont ou Halles et République. Je ne voudrais pas, enfin, que la ville de Tourcoing ...

Ce n'est pas une vue de l'esprit : c'est un vrai risque, avec des conséquences dommageables pour notre économie. Ainsi, permettez-moi de citer un autre exemple très concret : la Seine-Saint-Denis va accueillir les jeux Olympiques en 2024. de la gestion de nombreux parkings ? Des équipements à venir ? Des services tels que la gestion de l'eau ou des déchets ? Les associations d'élus locaux ont fait valoir également leurs préoccupations et se sont fait le relais auprès des ministres concernés, Jacqueline Gourault et Sébastien Lecornu. Je sais pouvoir compter sur l'écoute de ces derniers, car c'est bien le coeur même de l'action publique locale qui est concerné. N'oublions pas que les EPL constituent un prolongement de l'action des collectivités, et cette mobilisation traduit aussi l'attachement des élus à leur liberté d'action à un moment où la notion même de décentralisation est quelque peu malmenée. Jusqu'à présent, nous avons des outils qui fonctionnent, permettant la coopération entre strates locales, surtout dans un contexte où les EPL seront de plus en plus sollicitées avec la mise en oeuvre de la loi Élan. Je tiens à remercier l'ensemble des groupes parlementaires de cette assemblée qui ont bien voulu s'associer à ma démarche et la soutenir. Mes remerciements vont notamment, je le répète, à mes collègues Antoine Lefèvre, Julien Bargeton, Sylvie Robert, Alain Fouché et bien d'autres, qui ont cosigné cette proposition de loi.

comme si le soupçon devait en permanence peser sur les EPL et les élus. C'est d'autant plus cocasse que le Président de la République s'évertue depuis plusieurs semaines, à force de réunions-marathons, à renouer le fil du dialogue avec les élus locaux, en leur promettant de faciliter leurs actions. J'espère que cette proposition de loi, passé le cap sénatorial, saura trouver un écho favorable à l'Assemblée nationale. L'avenir nous le dira très rapidement. Je le répète, il était surtout urgent d'agir. Le législateur est dans son rôle pour préciser les conditions de fonctionnement des SPL et, par conséquent, pour rétablir une certaine forme de sérénité chez les acteurs locaux. La parole est à M. le rapporteur.

au Sénat, nous connaissons tous parfaitement la place prépondérante des entreprises publiques locales et de l'économie mixte à l'échelle de nos territoires. Ces sociétés de droit privé, dont le capital est totalement ou partiellement public, permettent de faire converger les moyens et les énergies pour conduire nombre de projets, qui concernent aussi bien l'aménagement, l'immobilier ou les services publics locaux. La Caisse des dépôts et consignations nous l'a confirmé : les sociétés publiques locales, les sociétés publiques locales d'aménagement-SPLA-et les sociétés d'économie mixte-SEM-locales sont des éléments clés du dynamisme de nos territoires. Leur succès rend aujourd'hui les EPL incontournables. Il en existe 1 300 en activité, dont plus de 900 SEM locales et plus de 350 sociétés publiques locales et sociétés publiques locales d'aménagement.

Mais ces sociétés courent aujourd'hui un danger grave. Par une décision du 14 novembre 2018, le Conseil d'État a imposé, de manière prétorienne, que chaque collectivité actionnaire détienne désormais l'ensemble des compétences sur lesquelles porte l'objet social de la société. D'un trait de plume, le juge administratif a plongé dans l'incertitude la très grande majorité des EPL existantes et bloqué la plupart des projets de création. Cette jurisprudence ne s'appliquait qu'aux seules SPL, mais les SPL d'aménagement et les SEM locales devraient également être concernées, puisqu'elles sont soumises à des dispositions similaires. Or la majorité de ces sociétés sont capitalisées par des collectivités ou des groupements de collectivités qui ne détiennent pas l'ensemble des compétences sur lesquelles porte l'objet même de ces sociétés. En l'état, cette jurisprudence sonne donc le glas des EPL « multicouches et de la coopération entre collectivités. Plus grave, une SPL ne peut exercer son activité que pour le compte des collectivités ou des groupements qui en sont actionnaires. Diminuer le nombre de collectivités pouvant participer au capital limite donc le nombre de « clients

Afin de rendre la proposition plus claire, la commission des lois a souhaité qu'elle n'introduise que des dispositions strictement nécessaires à la mise en échec de la jurisprudence du Conseil d'État, pour ne pas bouleverser inutilement le droit applicable. Nous avons également souhaité que la formulation retenue lève toute ambiguïté sur le rôle des entreprises publiques locales, qui sont des prestataires et non pas des EPCI. Sociétés commerciales strictement tenues par leur objet social, les entreprises publiques locales n'exercent aucune compétence en lieu et place des collectivités actionnaires. Elles fournissent des prestations, pour leur compte et sous leur contrôle, afin que celles-ci exercent leurs compétences. En ce qui concerne l'extension du champ de la proposition de loi, nous avons souhaité que celle-ci s'applique aussi aux SPL d'aménagement et aux SPL d'aménagement d'intérêt national. Cette extension est justifiée par la volonté

Enfin, l'article 4 de la proposition de loi a été introduit afin de valider l'actionnariat des entreprises publiques locales existantes qui ne respectent pas le nouveau critère fixé par le Conseil d'État. Nous aurons l'occasion de revenir sur ce point lors de l'examen des amendements. outre, la commission a déposé un amendement de séance tendant à fixer les modalités d'application outre-mer de cette proposition de loi. Pour faire obstacle à toute irrecevabilité financière, je dois vous demander, monsieur le secrétaire d'État, de bien vouloir donner votre accord à cette application ultramarine. Il s'agit d'un accord sur le principe, car les amendements déposés par le Gouvernement montrent que nous devons encore nous accorder sur un certain nombre de points. Comme je l'ai dit, nos territoires attendent une réponse rapide de notre part. Je pense, en revanche, que cette réponse ne doit pas être formulée au détriment de la clarté et de la prévisibilité du droit applicable aux entreprises publiques locales. Au cours de l'examen des amendements, je n'aurai de cesse de le rappeler. Nous ne devons pas

Monsieur le président, monsieur le président de la commission des lois, monsieur le rapporteur, monsieur le président Marseille, auteur de la proposition de loi, mesdames, messieurs les sénateurs, je souhaite tout d'abord excuser l'absence de Jacqueline Gourault, qui est aujourd'hui aux côtés du Président de la République en Corse, dans le cadre de la réunion qu'il organise avec les maires de l'île. Elle m'a demandé de la représenter, ce que j'ai accepté avec grand plaisir, pour l'examen de ce texte important pour les entreprises publiques locales et les collectivités territoriales. Le Gouvernement considère que l'initiative législative que vous avez prise, monsieur le président Marseille, est bienvenue dans le contexte de fortes contraintes juridiques, pour ne pas dire excessives, résultant de la récente décision du Conseil d'État, qui a été mentionnée à plusieurs reprises. Il est Il est en effet urgent d'améliorer le droit applicable à l'actionnariat des entreprises publiques locales, afin de ne pas prendre le risque de déstabiliser un secteur économique essentiel à la vie de nos territoires. Ce n'est pas à vous, mesdames, messieurs les sénateurs, que j'apprendrai à quel point ces entreprises jouent un rôle majeur dans la vie économique locale. Si l'on se réfère aux statistiques fournies par la Fédération des entreprises publiques locales, publiques locales, les collectivités ont créé près de 1 300 entreprises publiques locales, dont 925 sociétés d'économie mixte locales, 359 sociétés publiques locales et 16 sociétés d'économie mixte à opération unique. Ces entreprises emploient près de 70 000 salariés et représentent environ 14 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Au-delà de ce rappel purement statistique, il faut noter que le champ d'action des EPL s'est enrichi et a évolué avec la pratique. Ces entreprises constituent l'un des nombreux outils dont disposent les collectivités territoriales pour mener à bien leurs missions parmi une palette de possibilités. L'économie mixte contribue ainsi au dynamisme du développement territorial et au soutien de l'investissement local. C'est un mode d'action permettant de faire émerger des politiques innovantes, telle la transition énergétique. Ces

En outre, des secteurs comme l'habitat et l'immobilier ou la mobilité confirment leur importance, tandis qu'émergent de nouveaux champs d'action comme l'environnement, les réseaux, le développement économique et les services à la personne. À cet égard, il est intéressant de noter que certains domaines comme le tourisme, la culture, le sport et l'énergie renouvelable relèvent de compétences partagées entre différents niveaux de collectivités territoriales, ce qui nous amène directement au sujet dont nous débattons aujourd'hui. En effet, autrefois exceptionnelle, la pluriactivité des entreprises publiques locales est désormais majoritaire, ce qui rend d'autant plus nécessaires les adaptations juridiques auxquelles nous invite la décision du Conseil d'État du 14 novembre 2018. constant sur ce point : une collectivité n'a pas le droit de faire, par l'intermédiaire d'une société d'économie mixte locale ou d'une société publique locale, ce qu'elle n'a pas le droit de faire par elle-même. Cette règle, qui n'est d'ailleurs pas remise en cause par la proposition de loi, est du reste antérieure à la loi NOTRe, car elle date des premiers textes ayant instauré la possibilité de créer des entreprises publiques locales. Toutefois, la jurisprudence administrative hésitait jusqu'à présent entre deux interprétations pour ce qui concerne la situation des sociétés exerçant dans plusieurs champs d'activité. Selon l'interprétation la plus souple, une collectivité ne pouvait participer que si la part prépondérante des missions de la société n'outrepassait pas son domaine de compétence. Selon l'interprétation la plus stricte, une collectivité ne pouvait participer au capital d'une entreprise publique locale que si elle détenait la totalité des compétences correspondant aux missions de l'entreprise. C'est une lecture stricte de la loi que le Conseil d'État a retenue au mois de novembre dernier. On estime ainsi qu'un grand nombre d'entreprises locales, près de 40 % d'entre elles, ne rempliraient plus les conditions posées par la jurisprudence. Il était donc urgent de revenir sur cette jurisprudence, ce que prévoit opportunément cette proposition de loi. Le Gouvernement partage l'objectif poursuivi par les auteurs de ce texte, dont l'économie générale n'a pas été modifiée par la commission des lois, puisque le rapporteur, dont je salue le travail, a apporté des compléments utiles, en particulier en étendant expressément les dispositions du texte aux sociétés publiques locales d'aménagement. Toutefois, je souhaite dire dès ce stade de notre discussion que le Gouvernement craint que la rédaction retenue par la commission des lois ne constitue un assouplissement excessif de la législation en vigueur. Il s'agit non pas de soupçons, monsieur le président Marseille, mais plutôt de précautions. Ainsi, le texte résultant des travaux de la commission des lois n'interdirait pas à une collectivité de prendre une participation élevée dans le capital d'une entreprise publique locale, quand bien même les activités de cette dernière ne correspondraient que pour une part très marginale à des compétences exercées par cette même collectivité. Au surplus, il nous semble que cette même rédaction ne fait pas clairement obstacle à ce qu'une partie de l'activité de l'EPL ne relève d'aucune compétence des collectivités actionnaires. Nous craignons qu'un tel choix ne permette, d'une part, de régulariser des SPL et sociétés d'économie mixte locales qui étaient déjà non conformes avec le droit antérieur à la décision du Conseil d'État et, d'autre part, d'encourager le recours à des entreprises publiques locales à objets sociaux multiples,

notre analyse, réel. Le Gouvernement souhaite par conséquent que le droit permette de limiter le risque de voir des collectivités investir des missions ne relevant pas de leur champ de compétence. Ce raisonnement nous a conduits à déposer des amendements aux articles 1, 2 et 3 de la proposition de loi visant à encadrer la possibilité, pour les collectivités et leurs groupements, de prise de participation au capital d'une EPL dans des conditions plus resserrées, en prévoyant qu'une telle participation ne soit possible que si la collectivité ou le groupement ne détient pas au moins une compétence sur laquelle porte l'objet social de la société et à laquelle celle-ci consacre une part significative et régulière de son activité.

qu'une telle précision est indispensable. Je ne m'attarderai pas sur ce point à ce stade du débat, puisque nous aurons l'occasion d'y revenir à l'occasion de l'examen des amendements. Je voudrais, pour conclure, dire que le débat d'aujourd'hui doit également nous conduire, selon l'analyse qu'en fait le Gouvernement, à nous pencher sur la régulation du secteur des entreprises publiques locales. En 2017, deux études ont porté sur les entreprises publiques locales : un référé de la Cour des comptes sur le cadre juridique et comptable applicable, ainsi qu'une revue de dépenses des inspections générales sur la maîtrise des risques par les EPL. Ces deux rapports, rendus publics, se sont avérés très critiques, leurs auteurs plaidant en faveur d'un renforcement du contrôle des EPL et de leurs filiales. Dans son référé du 15 juin 2017, la Cour des comptes a notamment fait valoir que les EPL, instruments essentiels pour les collectivités, ne sont pas « suffisamment maîtrisés » et que « les mécanismes de leur contrôle, de leur transparence et d'évaluation de leur contribution à l'action publique territoriale devraient être repensés ». Les conclusions d'une nouvelle étude de la Cour des comptes sur le même sujet, conduite à la demande du président de la commission des finances de l'Assemblée nationale, nationale, sont d'ailleurs attendues dans les prochaines semaines. À ma connaissance, ce rapport devrait aussi être rendu public. Dans ces conditions, le Gouvernement estime que le législateur pourrait se saisir de ce débat pour apporter une réponse, en concertation avec les représentants des collectivités territoriales et des entreprises publiques locales, à ces remarques émises par la Cour des comptes. constituerait à l'évidence un facteur d'équilibre et de sécurisation de l'activité des entreprises publiques locales, en complément des assouplissements proposés par le texte dont nous débattons aujourd'hui. Mesdames, messieurs les sénateurs, je souhaite pour finir remercier de nouveau les auteurs de ce texte pour leur initiative et vous assurer de l'ouverture d'esprit du Gouvernement. La discussion d'aujourd'hui doit nous permettre de parvenir à une solution équilibrée, dans le respect des différentes contraintes juridiques que je viens de rappeler. Je ne doute pas que la poursuite de l'examen de ce texte par l'Assemblée nationale, puis dans le cadre de la navette parlementaire, nous permettra d'atteindre un point d'équilibre satisfaisant pour chacune des parties. La parole est

l'administration centrale est toujours extrêmement méfiante à l'égard des collectivités locales et n'a pas compris, depuis 1983, l'intérêt des sociétés d'économie mixte ni, depuis 2010, celui des sociétés publiques locales.

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, à l'heure où l'on demande à nos collectivités de faire toujours plus d'économies, d'être toujours plus innovantes, les entreprises publiques locales sont bien souvent un outil de développement et de mutualisation incontournable.

Les membres du RDSE, par les voix d'Anne-Marie Escoffier et de Jacques Mézard, avaient alors pris leur part dans la proposition de loi qui avait été à l'époque adoptée à l'unanimité des deux chambres. La proposition de loi dont nous débattons aujourd'hui, par la souplesse qu'elle permet de redonner à notre économie locale, repose sur un large consensus. Je tiens d'ailleurs à remercier notre collègue Loïc Hervé

d'exercer l'ensemble des compétences sur lesquelles porte l'objet social de ladite société, assimile les EPL aux EPCI, créant ainsi une grande insécurité pour les 1 300 entreprises publiques locales dont, en France, nous disposons et gelant les projets en cours de création insécurité juridique concernant la légalité des actes des SPL existantes qui ne répondraient pas au nouveau critère défini par le Conseil d'État ; risque d'émiettement et de dilution de l'action publique locale pour les SPL en cours de création, qui verraient leurs projets mis à l'arrêt. Au-delà de ces considérations juridiques, l'entérinement de cette décision viendrait plonger les EPL et nos collectivités dans une insécurité économique. On mettrait fin aux efforts de mutualisation et aux économies de gestion qu'a permis la création de nombreuses SPL. On réduirait le nombre de collectivités

porte atteinte aux projets locaux et à l'apport des entreprises publiques locales au dynamisme de nos territoires. Nous le voyons tous : à l'échelle locale, nos EPL rendent possible le lancement de projets à long terme, dans des domaines comme le tourisme, la culture ou l'aménagement. Elles sont le fer de lance de l'investissement et de l'innovation sur nos territoires et participent également à leur revitalisation. Dans les territoires touristiques, elles permettent une souplesse commerciale plus importante qu'en régie, les élus se retrouvent confrontés à une lourdeur administrative qui les oblige parfois à délibérer sur le moindre petit acte commercial. Les SEM ou les SPL donnent une souplesse d'action et de réaction tout en préservant la maîtrise de la collectivité et la transparence de ses comptes, n'en déplaise à l'administration. Les conseils départementaux, ayant perdu la clause générale de compétence avec la loi NOTRe, se verraient aujourd'hui privés également d'un grand nombre d'outils locaux indispensables à l'avenir de leurs territoires. Dans un département comme les Hautes-Pyrénées, où les collectivités sont obligées de pallier une initiative privée frileuse ou manquante dans des domaines essentiels à la vie économique de notre territoire, comme le thermalisme ou les sports d'hiver, ces organisations sont aujourd'hui nombreuses et confrontées au redécoupage territorial des communautés de communes et aux redéfinitions de compétences correspondantes. Ces outils nouveaux ont démontré qu'ils pouvaient être de vraies réussites, en témoigne l'exemple de la SEM N'Py, pour « Nouvelles Pyrénées », qui, regroupant les huit principales stations de ski pyrénéennes, permet de mener une stratégie commerciale offensive et de mutualiser certains outils, donc de rationaliser les coûts de fonctionnement. Pour en revenir au texte qui nous est présenté, la décision du 14 novembre est un non-sens unique en Europe. On considère les SPL comme des EPCI, alors que leur succès repose sur cette différentiation commission, qui précise que la réalisation de l'objet de la société concourt à l'exercice d'au moins une compétence de chacun des actionnaires, permet de rétablir la souplesse

localement. Dans l'esprit qui le caractérise, le groupe du RDSE votera à l'unanimité pour ce texte d'une importance capitale pour le dynamisme de nos territoires. La parole

Marseille. Elle remédie à une jurisprudence du Conseil d'État qui conçoit de façon restrictive le lien de compatibilité entre les compétences des actionnaires et l'objet d'une société publique locale. Le 14 novembre dernier, le Conseil d'État a opté pour une lecture rigoriste de l'article L. 1531-1 du code général des collectivités territoriales. Aux termes de cet article, les collectivités et leurs groupements peuvent créer des sociétés publiques locales dans le cadre des compétences qui leur sont attribuées par la loi. à une société publique locale est exclue lorsque cette collectivité ou ce groupement n'exerce pas l'ensemble des compétences sur lesquelles porte l'objet social de la société. La participation au capital d'une telle société confère la qualité d'actionnaire et ouvre donc le droit de participer au vote des décisions prises par la société. Adopter une lecture moins rigoriste du texte permettrait à une collectivité de voter sur des sujets échappant à sa compétence, et donc d'exercer une compétence qu'elle n'a pas. Le Conseil d'État a estimé qu'il ne disposait d'aucune base légale pour autoriser Cette jurisprudence limite dangereusement la liberté d'action des collectivités et de leurs groupements. Elle impose l'intervention du législateur. Son application remet en cause la légalité des actes des sociétés publiques locales irrégulièrement composées.

Cette jurisprudence présente également un risque économique, puisque les sociétés publiques locales ne peuvent exercer leur activité qu'au profit des collectivités ou groupements qui en sont actionnaires. Restreindre le nombre de collectivités ou de groupements pouvant être actionnaires revient à restreindre les « clients » potentiels de ces sociétés, ce qui aura un effet négatif sur leur chiffre d'affaires. Les entreprises publiques locales sont des éléments clés du dynamisme de nos territoires. Elles représentent 65 000 emplois, 14 milliards d'euros de chiffre d'affaires et fournissent un logement à 1,4 million de personnes en France. Elles contribuent à la cohésion et au développement des territoires en matière d'innovation économique, de logement social, d'énergies renouvelables, de mobilité, d'attractivité touristique ou de revitalisation des coeurs de ville. Notre collègue Hervé Marseille a cité les villes du nord

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, j'aimerais tout d'abord saluer la convergence de vues sur les différentes travées de cet hémicycle, puisque la présente proposition de loi a été cosignée par des membres de six des sept groupes que compte notre assemblée, dont votre serviteur. Ce fait est suffisamment original pour être souligné, et je veux parier que nos collègues du groupe CRCE nous rejoindront pour un vote positif. Ce qui explique notamment ce consensus, c'est l'expérience des parlementaires qui, jadis, ont souvent été maires ou présidents de collectivité, n'en déplaise à certains, et qui, dans le cadre de la gestion quotidienne de leur collectivité, ont pu mesurer combien il était nécessaire de moderniser régulièrement le statut des SEM.

ailleurs rappeler le principe majeur qui est au fondement de la décentralisation, principe que le Conseil constitutionnel s'efforce, vaille que vaille, texte après texte, de faire respecter : celui de la liberté laissée à toute collectivité territoriale, petite ou grande, commune, département, région ou nouvelle communauté, pour réaliser ses interventions. Les chamboulements des dernières années en matière de regroupements ont durablement transformé le paysage de la France. Les 1 300 sociétés d'économie mixte sont, dans notre paysage institutionnel et dans la pratique de la gestion des collectivités locales, une réalité qui a pris beaucoup d'importance, même si, leur origine étant lointaine-les décrets-lois Poincaré datent de 1926-, la progression en a été étalée dans le temps. L'histoire des entreprises publiques locales s'est toujours faite par les élus, et le Parlement s'est régulièrement saisi de textes les instaurant, les remaniant, les aménageant, les actualisant, du fait des nouvelles responsabilités que les collectivités locales doivent, et devront, assumer. Les EPL sont des outils créés par les élus pour leur territoire, et dont ils ont la maîtrise politique et financière. Le montant de leur capitalisation s'élève à 4,3 milliards d'euros, détenus à 65 % par les collectivités locales ; autrement dit, elles représentent une opportunité de développement inouïe. Le rôle des parlementaires est donc important dans leur histoire récente, et nous sommes très sensibles à la question de leur sécurité juridique. Chaque texte de loi relatif aux entreprises publiques locales, ou presque, a été voté à l'unanimité-cela a été rappelé.

notre collègue Hervé Marseille, que je remercie de nouveau, et par notre rapporteur, vise donc à sécuriser les SEM et les SPL, si indispensables à nos territoires, en permettant aux collectivités locales de différents niveaux d'en être actionnaires.

grand comique ! Nul doute que l'arrêt du 14 novembre 2018 a été d'une redoutable efficacité en matière d'incitation-les précédents orateurs ont dit combien l'émotion et l'inquiétude étaient fortes dans leur territoire. été très heureux, après avoir été sollicité notamment par le président de la communauté d'agglomération de Marne et Gondoire, au moment où je commençais à travailler sur le sujet, de constater qu'Hervé Marseille avait fait preuve d'une diligence tout à fait inouïe, diligence ... ... qu'on lui connaît ! ... qui le caractérise, en prenant l'initiative de cette

n'aborde plus les SPL comme un outil au service des actionnaires, mais comme leur prolongement organique. Dès lors, par son considérant de principe, le juge de cassation estime que « la participation d'une collectivité est exclue lorsque cette collectivité n'exerce pas l'ensemble des compétences sur lesquelles porte l'objet social de la société ». Il faut donc l'arbitrage du législateur. Oui ! Ce n'est pas une question de « défiance », pour reprendre le mot de Jacques Bigot : il appartient bien au législateur d'intervenir. J'ai d'ailleurs constaté, dans les précédentes interventions, un accord

La commission des lois-c'est mon second point-a souhaité apporter quelques éléments de clarification rédactionnelle et étendre le champ d'application du texte aux SPLA, ce qui est certainement très bien. Le seul désaccord, marginal,

Je n'ai pas la prétention de penser que cet amendement puisse servir de compromis utile pour répondre aux observations du Gouvernement sans détricoter le travail consensuel de la commission des lois, mais nous avons vraiment, me

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, je ne rappellerai pas l'importance prise par les SPL dans la vie de nos collectivités-cela a été fait, et bien fait. Pour moi, les choses sont très claires : on ne peut que soutenir le texte de notre commission, un texte qui rétablit la portée de la loi initiale sur les SPL, soigneusement obscurcie et limitée par la jurisprudence administrative. Je n'en suis d'ailleurs pas surpris ; à ceux qui le seraient, je conseille la lecture du rapport du Conseil d'État de 2002 sur les collectivités publiques et la concurrence. Je cite La promotion du service public commence dans une pleine reconnaissance du cadre d'ensemble de libre concurrence dans lequel il est appelé à intervenir.

pour conclure, que, si j'avais encore quelques doutes sur l'intérêt du texte présenté par la commission, les amendements clairement restrictifs, eux aussi, du Gouvernement, les lèveraient. Mais nous aurons l'occasion d'y revenir.

a souligné que la position du Conseil d'État pouvait avoir des « effets dévastateurs pour l'action des entreprises publiques locales » et porter « une atteinte immédiate à la viabilité économique d'un grand nombre de SPL ». L'effet serait

C'est donc de manière parfaitement assumée que l'article 1 de la proposition de loi remet expressément en cause la jurisprudence du Conseil d'État, qui impose que toutes les compétences soient détenues

un objet simple et précis : elle vise à sécuriser définitivement le régime juridique des entreprises publiques locales, et non à introduire des dispositions qui pourraient nourrir une jurisprudence abondante. Notre rapporteur a parfaitement compris cet objectif.

elle ne vise rien de moins que la sauvegarde et la pérennisation des EPL. Je ne reviendrai pas sur l'analyse de l'arrêt du Conseil d'État. La proposition de loi vient vraiment clarifier et sécuriser juridiquement le paysage des EPL, en restant fidèle à la lettre de la loi de 2010 et en prenant en considération les évolutions observées en France, mais aussi en Europe, ces outils au service de la décentralisation. Plus précisément, elle fixe le principe suivant : la réalisation de l'objet de l'EPL doit « concourir à l'exercice d'au moins une compétence de chacun des actionnaires ». En somme, il s'agit de faire preuve de souplesse, de cohérence, mais aussi d'efficacité. Affaiblir et limiter le recours aux EPL va à l'encontre du contexte actuel, qui favorise au contraire l'appel à ces structures par les collectivités. Trois facteurs en particulier vont dans ce sens. Premièrement, le tarissement des dotations de l'État aux collectivités

qui semblent le mieux adaptées à cet environnement en pleine mutation. Les EPL représentent justement une de ces modalités. Deuxièmement, les EPL s'inscrivent dans une conception moderne de l'action publique, fondée sur une logique partenariale et de projet territorial. Il s'agit bien de créer, à l'échelle d'un territoire, les synergies nécessaires entre acteurs publics ou entre acteurs publics et privés en vue de l'accomplissement d'une mission d'intérêt général. Dans ce cadre, des mutualisations peuvent être opérées, les savoir-faire peuvent être partagés et, d'une manière générale, la gestion est efficiente. Troisièmement, les EPL peuvent vraiment, à mon ce nouveau mouvement de décentralisation que beaucoup appellent de leurs voeux. La tendance à vouloir renforcer l'action publique de proximité et à ancrer territorialement les politiques publiques stimule l'essor des EPL. En 2018, leur nombre s'est accru de 4 %, et leurs activités se sont diversifiées ; je pense notamment aux domaines de la culture et du tourisme.

les EPL peuvent être utiles au rééquilibrage économique, social et culturel entre les territoires. Dans le contexte actuel, ce n'est pas anodin.

Mme Christine Lavarde. « Le Conseil d'État a encore frappé avec un manque total de nuances. » C'est en ces termes qu'Éric Landot, avocat à la Cour, a commenté le fameux arrêt rendu par le Conseil d'État le 14 novembre dernier. Les SPL ont été créées en 2010 pour donner aux collectivités territoriales la souplesse des entreprises privées tout en garantissant un contrôle complet par les actionnaires publics. En effet, à la différence des SEM, elles ne comptent pas d'actionnaires privés à leur capital. Cette souplesse, si rare en matière de commande publique, a été très appréciée des collectivités territoriales. De nombreuses SPL ont vu le jour depuis 2010 dans des domaines divers : aménagement de centre-ville, assainissement, déploiement du numérique jours après la publication de l'arrêt du Conseil d'État, d'application immédiate, le préfet des Hauts-de-Seine adressait à l'ensemble des collectivités du département le courrier suivant : « [ ...] S'il était établi qu'une collectivité ne pouvait être actionnaire d'une SEML ou d'une SPL dès lors qu'aucune de ses compétences ne figurait dans les statuts de la société, restait à trancher le cas des sociétés à " objet mixte ", dont les missions ne relèvent qu'en partie de la compétence de la collectivité. [ ...]. Dans un arrêt du 14 novembre 2018, le Conseil d'État retient la lecture selon laquelle toutes les missions de la société doivent relever de la compétence de la collectivité. Aussi, je vous invite, lorsque votre collectivité ou votre établissement se trouve dans ce cas de figure, à engager, dans les meilleurs délais, les cessions d'actions qui s'imposent au sein des SEM et des SPL dont les missions ne correspondent pas intégralement à ses compétences Faire évoluer l'actionnariat des SPL est plus complexe que ne le laisse apparaître ce courrier. Les SPL ne peuvent compter ni sur l'actionnariat public national ni sur l'actionnariat privé pour remplacer les actionnaires ne disposant pas d'une identité de compétence. Or une SPL ne peut exister en l'absence de deux actionnaires publics locaux.

Au-delà de la potentielle difficulté à trouver un nouvel actionnaire prêt à acquérir les parts cédées, qui pourrait imaginer qu'une commune du périmètre de la métropole du Grand Paris ayant acquis sur ses fonds propres un terrain en friche devienne un actionnaire très minoritaire de la SPL qui l'aménage ? C'est l'ex-administratrice de la SPL Val de Seine Aménagement, qui porte le projet emblématique de l'île Seguin, qui vous parle pour sécuriser l'ensemble des opérations et des contrats en cours gérés par les 169 SPL et les 333 SEM, recensées par la rapporteure publique du Conseil d'État, dont l'objet social excède le champ des compétences partagées par leurs actionnaires, il y a urgence à venir préciser l'esprit de la loi et la volonté et la volonté du législateur. Au-delà de ce texte, qui vient régler une difficulté précise-je profite de l'occasion pour remercier mon voisin, le président Hervé Marseille, de son initiative-, je ne peux qu'inviter le Gouvernement, qui s'est montré si frileux jusqu'ici, notamment lors du congrès des EPL à Rennes au mois de décembre dernier, à ouvrir un débat juridique sur la réglementation des sociétés publiques locales, outil indispensable à l'aménagement de nos territoires. La décision du Conseil d'État risque fort de faire jurisprudence pour les SPLA. Il conviendrait donc de modifier également les dispositions de l'article L. 327-2 du code de l'urbanisme La réflexion pourrait également s'engager sur la manière dont la France pourrait appliquer les règles plus souples de l'Union européenne en matière de, sans systématiquement sur-transposer.

de la réglementation, en encourageant le recours à des entreprises publiques locales à objets sociaux multiples, alors même que la compétence de la collectivité ne correspondrait qu'à une part négligeable des activités de la société. Par ailleurs, selon nous, la rédaction proposée ne fait pas clairement obstacle à ce qu'une partie de l'activité de la SPL ne relève d'aucune des compétences des collectivités territoriales ou des groupements actionnaires. En effet, la formulation

Si la compétence des collectivités territoriales ne se confond pas avec l'objet social de la société, celui-ci doit être défini de manière précise, afin que le lien avec les compétences des collectivités ou groupements actionnaires puisse être clairement établi, comme le rappelle la circulaire du 29 avril 2011 relative au régime juridique des sociétés publiques locales. Par conséquent, cet amendement a pour objet de préciser que les collectivités et leurs groupements ne peuvent être actionnaires d'une société publique locale s'ils ne détiennent pas au moins une compétence sur laquelle porte l'objet social de cette dernière. Cette compétence doit en outre correspondre à une « part significative et régulière » de l'activité de la société.

De plus, la formule proposée nous paraît plus souple que la fixation dans la loi d'un seuil chiffré, dont l'application ne manquerait pas de créer de nombreuses difficultés. Pour ces raisons, je vous demande de bien vouloir adopter cet amendement.

Qu'est-ce qu'une « part » d'activité ? À partir de quand est-elle « significative » ? Comment mesurer si elle est « régulière » ? Je ne le sais pas, et c'est probablement au juge

Derrière l'utilisation de ces critères flous se cacherait en réalité le recours au bon vouloir des préfets. Ils disposeraient d'un droit de vie ou de mort sur les projets d'EPL, pouvant brandir la menace d'un contentieux tout à fait aléatoire. L'utilisation du critère de la régularité leur permettrait même de remettre en cause l'existence d'EPL déjà constituées. C'est d'ailleurs ce qui se passe actuellement dans un certain nombre de départements : des entreprises publiques locales reçoivent des courriers des préfets. L'insécurité juridique manifeste qui découlerait d'une telle rédaction porterait préjudice aux entreprises publiques locales, aux collectivités qui en sont actionnaires et,, aux projets et à la population des territoires concernés.

Cette mention fait donc obstacle à ce que des collectivités ou groupements créent des entreprises publiques locales dont la réalisation de l'objet concourrait à l'exercice de compétences qu'ils n'ont pas.

la commission, précise que les dispositions du texte s'appliquent aux sociétés constituées antérieurement à sa publication. Nous estimons que l'utilité de cette mesure n'est pas démontrée, dès lors que les dispositions de la loi ont vocation à s'appliquer à toutes les sociétés à compter de sa publication. Par ailleurs, le Conseil constitutionnel contrôle de manière stricte les validations législatives, sur le fondement du respect des cinq conditions suivantes : la validation doit être justifiée par un motif impérieux d'intérêt général ; elle doit respecter les décisions de justice ayant force de chose jugée doit respecter le principe de non-rétroactivité des peines et des sanctions ; l'acte validé ne doit méconnaître aucune règle ni aucun principe de valeur constitutionnelle, sauf à ce que le but d'intérêt général visé par la validation soit lui-même de valeur constitutionnelle

À l'exception des dispositions d'ordre public, le droit qui leur est applicable est donc celui qui était en vigueur au moment de leur conclusion. En conséquence, si nous voulons que les dispositions que nous examinons s'appliquent aux EPL existantes, il faut explicitement le prévoir en les validant. C'est précisément la raison d'être de l'article 4, qui est donc parfaitement nécessaire. Les entreprises publiques locales existantes représentent près de 14 milliards d'euros de chiffre d'affaires

Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, madame la rapporteure, mes chers collègues, nous avons terminé l'année 2018 par des célébrations en l'honneur des soldats tombés pour la France et des millions de morts causés par la Première Guerre mondiale. Le Président de la République a effectué une itinérance mémorielle dans les départements de l'Est et du Nord, qui ont payé un lourd tribut au cours de la Grande Guerre. Des honneurs ont été rendus aux combattants, tant pays que chez nos amis étrangers ; de nombreux pays avaient envoyé leurs enfants combattre aux côtés des Français lors de la guerre de 14-18. Mon département, la Marne, situé au centre des conflits armés des deux guerres mondiales, était, bien entendu, au coeur des commémorations depuis quatre ans déjà. Les pouvoirs publics, les établissements scolaires, les collectivités locales, les associations culturelles ou celles des anciens combattants se sont mobilisés pour le centenaire de la fin de la Grande Guerre, au travers de cérémonies commémoratives, de spectacles, de lectures, de débats ou de chorales. Les médias français se sont mobilisés pour rendre compte de l'indispensable travail mémoriel. Ceux du monde entier se sont massivement déplacés pour assister aux vibrantes cérémonies du 11 novembre Hymnes nationaux scandés par les enfants, reconstitutions historiques en tenues militaires des différents pays, défilés patriotiques guidés par la fanfare ... et les porte-drapeaux Une cérémonie commémorative n'aurait pas la même portée symbolique sans les trois couleurs hissées aux bras des anciens combattants et des bénévoles animés par le devoir de mémoire. Chacun d'entre nous salue ces hommes, ces femmes qui arpentent les rues de nos villages et de nos villes, souvent plusieurs fois dans la journée, sous la pluie, le vent, la neige ou la canicule pour un périple historique, solennel, en hommage aux morts pour la France. Chaque drapeau tricolore siglé de l'acronyme d'une association reflète une part de l'histoire de France. Chaque pavillon bleu-blanc-rouge évoque fièrement les épreuves dures et intenses traversées 14-18, 39-45, Algérie, Indochine, Afghanistan, Mali ... Je ne pourrai malheureusement toutes les citer, cette liste n'ayant, hélas, pas de fin. Ces drapeaux colorent nos défilés et font la fierté des enfants qui assistent aux cérémonies.

celle de faire partie de la même patrie, de se souvenir de ces valeureux jeunes enrôlés dans la défense de la liberté de leur pays et des valeurs auxquelles ils croyaient.

En effet, les porte-drapeaux et les responsables des associations vieillissant, les sections locales disparaissent progressivement. La plupart des drapeaux trouvent refuge dans une autre association, entre les mains d'un autre bénévole perpétuant la mémoire au pied du monument aux morts et des stèles commémoratives, certains d'entre eux se retrouvent malheureusement dans des brocantes ou en vente sur des sites en ligne. L'alerte m'a été donnée par des anciens combattants, lors d'assemblées générales de sections locales ; certains d'entre vous ont fait le même constat dans leur département, et me l'ont rapporté. Les organismes représentatifs des anciens combattants et du souvenir m'ont relaté des faits similaires dans toute la France ; ils se trouvent démunis face à ces situations. Un drapeau tricolore est un objet commun que l'on peut acheter très simplement dans des magasins spécialisés ou sur internet ; tant mieux pour le patriotisme ! En revanche, un drapeau d'une association d'anciens combattants n'est pas un bien quelconque il est porteur de symboles, de valeurs, de respect pour nos aînés et l'histoire de France, ainsi que d'une forte empreinte historique et, bien souvent, sentimentale. Je remercie les plus de cinquante cosignataires du texte, siégeant dans différents groupes politiques, d'avoir contribué à l'émergence de cette discussion aujourd'hui. Leur large soutien va, sans conteste, droit au coeur des bénévoles et des porte-drapeaux. Des courriers de remerciement m'ont ainsi été adressés dès l'enregistrement de la proposition de loi à la présidence, en février 2018. Cela montre aux soldats et aux victimes que nous ne les oublions pas. J'ai voulu simplement retranscrire, au travers de ce texte, notre volonté de protéger les drapeaux des associations d'anciens combattants, qui sont une part de notre patrimoine commun.

Nous avons reformulé une partie du texte pour lever les doutes juridiques et garantir dans le temps la force de cette protection. Les membres de la commission présidée par Alain Milon ont entendu les arguments de la rapporteure et ont adopté, à l'unanimité, les modifications que nous nous étions attelées à parfaire conjointement, dans l'intérêt de la sauvegarde des emblèmes mémoriels. Chers collègues, il vous est proposé de considérer que le drapeau est un bien collectif, qui doit demeurer visible du grand public. Il ne doit pas être oublié dans un grenier ; il ne doit pas être mis aux enchères sur les sites de vente en ligne ; il ne doit pas être un vulgaire souvenir. Il est dans la mémoire collective ; il est notre patrimoine national Ainsi, il est proposé d'inscrire dans le droit qu'un drapeau portant les signes distinctifs d'une association d'anciens combattants est présumé, sauf preuve du contraire, appartenir à cette association. La prescription acquisitive ne pourrait ainsi plus être évoquée par la personne qui, ayant acquis d'une manière ou d'une autre un drapeau identifié comme appartenant à une association d'anciens combattants, revendiquerait en être le propriétaire légitime. Les associations pourraient par ailleurs obtenir gratuitement la restitution d'un drapeau leur appartenant qui aurait été vendu à l'occasion d'une brocante ou sur internet.

à moins que ses statuts ou son assemblée générale ne prévoient autre chose, il semble pertinent que ses biens-non seulement ses drapeaux, mais aussi, par exemple, ses archives-soient transférés à la commune de domiciliation. Celle-ci pourra les confier à des établissements scolaires, mais également à des musées ou à des fondations dont l'objet est la transmission de la mémoire, ou à toute autre structure qu'elle jugerait apte à perpétuer le travail mémoriel. Pour information, sachez que, lors de l'année scolaire 2017-2018, plus de 300 projets, portés par autant d'établissements scolaires, ont reçu le label « Centenaire » de la part de la mission du Centenaire ; cela témoigne de l'implication des jeunes et de leurs enseignants pour faire vivre le souvenir de la Grande Guerre. Le devoir de mémoire doit notamment passer par les jeunes générations. Il faut que ces drapeaux soient des outils pédagogiques pour l'apprentissage de la citoyenneté. Comme cela a déjà pu être expérimenté dans des lycées ou des écoles, un accord pourra être signé avec la mairie. le drapeau « reprendra vie » et pourra être porté par une classe, par exemple lors des cérémonies du 11 novembre ou du 8 mai. Le Sénat, représentant des collectivités locales, fait évidemment confiance aux communes pour organiser la transmission du souvenir au travers des drapeaux.

dont certains m'ont demandé comment agir, comment lutter contre cette dilapidation patrimoniale. Les organismes représentatifs que j'ai sollicités se trouvaient également démunis face à ce vide juridique. Il est heureux qu'un groupe de travail soit réuni par le ministère pour traiter des questions relatives aux objets militaires et de guerre dans leur ensemble. Des constats de revente ou de tentative de revente de plaques funéraires de combattants se sont fait jour au cours des dernières semaines.

Comment pourrions-nous évoquer la mémoire de nos grands-pères, tout en sachant que le drapeau qu'ils ont si fièrement porté se retrouve en vente sur internet ? Ces drapeaux sont les témoins du passé ; ils nous permettent de mesurer le prix de la liberté. Des hommes ont été tués, mutilés, blessés, choqués à vie en défendant notre liberté ou celle d'autres peuples. Mes chers collègues, rendons hommage à nos anciens ! Défendons leurs drapeaux ! Adoptons ce texte ! La parole

Alors que la première génération du feu, celle de la Première Guerre mondiale, a disparu, et que s'éteignent progressivement les anciens combattants de la deuxième génération, et même ceux de la troisième, qui ont combattu durant la Seconde Guerre mondiale, en Indochine ou en Afrique du Nord, la question de la transmission de la mémoire aux jeunes générations apparaît plus que jamais d'actualité. Chacun ici le sait pour le vivre sur son territoire : les associations d'anciens combattants jouent un rôle essentiel dans la politique mémorielle en assurant régulièrement les commémorations patriotiques qui rythment la vie de nos communes. Compte tenu de l'âge de leurs membres, ces associations ont malheureusement tendance à disparaître. Il arrive donc que leurs drapeaux soient oubliés, délaissés dans une cave ou un grenier. Il arrive également qu'ils soient mis en vente, par exemple par les héritiers d'un ancien combattant, d'un porte-drapeau, que ce soit sur internet ou lors de vide-greniers ou de brocantes, ce qui peut évidemment choquer. Le drapeau tricolore, que l'article 2 de la Constitution érige en emblème national, fait, depuis une date relativement récente, l'objet d'une protection juridique. L'outrage au drapeau constitue ainsi, selon les circonstances dans lesquelles il est commis, une contravention ou un délit, dont la punition peut aller jusqu'à trois ans d'emprisonnement. Toutefois, cette protection concerne le symbole que le drapeau représente et non l'objet lui-même, qui est, du point de vue du droit, un bien matériel privé. Malgré leur dimension patriotique et symbolique, les drapeaux appartenant ou ayant appartenu à des associations d'anciens combattants ne font pas exception. Au demeurant, ils sont librement acquis dans le commerce par ces associations. les acheteurs de ces drapeaux ne sont pas nécessairement mal intentionnés. Il s'agit souvent de collectionneurs passionnés d'histoire qui entendent traiter ces objets avec respect. Pour autant, aux yeux de certains de nos compatriotes, assimiler les drapeaux d'associations d'anciens combattants à des antiquités ordinaires conduit à nier leur dimension symbolique.

qui y voient un manque de considération de la société pour les services qu'ils ont rendus à la Nation et qui craignent que le souvenir qu'ils entretiennent au moyen de ces drapeaux ne s'efface. s'efface. Devant ce constat, l'auteur de la proposition de loi a souhaité garantir une protection des drapeaux appartenant ou ayant appartenu à des associations d'anciens combattants. Cet objectif est partagé par la commission des affaires sociales, qui a toutefois, sur ma proposition, amendé le texte initial afin de lever des difficultés juridiques qu'il posait, notamment pour écarter tout risque d'atteinte au droit constitutionnel de la propriété privée. Dans sa rédaction issue des travaux de la commission, la proposition de loi aménage le régime juridique de la prescription acquisitive, qui permet à un particulier de devenir légalement propriétaire d'un bien se trouvant en sa possession depuis un certain temps. Cette prescription ne serait ainsi plus applicable aux drapeaux appartenant à des associations d'anciens combattants, qui seraient présumés être la propriété de l'association dont ils portent les insignes, quand bien même ils auraient passé plusieurs années dans un grenier. En outre, une association pourrait obtenir gratuitement la restitution d'un drapeau lui appartenant qui aurait été indûment vendu sur un marché, sans avoir à rembourser l'acquéreur. Ces exceptions au droit commun sont apparues justifiées à la commission des affaires sociales, eu égard au caractère symbolique et patriotique des drapeaux en question et à la nécessité d'éviter que la disparition de nombreuses associations n'entraîne leur dispersion. Cette mesure devra s'accompagner d'une réflexion approfondie sur la perpétuation de la mémoire combattante, et je sais, madame la secrétaire d'État, que vous avez pris l'initiative de former un groupe de travail sur cette thématique. Voilà un peu moins d'un an, le Sénat examinait une proposition de loi relative à l'attribution de la carte du combattant aux soldats ayant servi en Algérie entre 1962 et 1964. Cette proposition de loi a été, pour le Gouvernement, l'occasion d'annoncer sur ce point précis une avancée depuis longtemps attendue par le monde combattant. Je forme donc le voeu qu'une fois encore l'initiative du Sénat joue un rôle d'aiguillon pour l'action gouvernementale. La commission des affaires sociales ayant adopté cette proposition de loi à l'unanimité, j'ose espérer qu'un même consensus émergera dans l'hémicycle cet après-midi. La parole

Monsieur le président, madame la rapporteure, mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs,

de nos mairies, de nos bâtiments officiels, au balcon de certains particuliers, dans la liesse populaire comme dans les heures de drame, ce drapeau est notre symbole de ralliement. de ralliement. Mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs, « le drapeau tricolore a fait le tour du monde avec le nom, la gloire et la liberté de la patrie » : c'est ce que disait en 1848 Alphonse de Lamartine, le grand poète national et républicain. Cela est toujours valable aujourd'hui. Sous ce drapeau, des femmes et des hommes ont porté l'uniforme, ont affronté le feu et sont morts pour la France. Ils l'ont fait en 1914, en 1940, en Indochine, en Algérie, dans nos opérations extérieures. Nos soldats le font encore avec dévouement et courage au Levant, au Sahel et dans d'autres endroits du monde.

Les drapeaux d'associations combattantes et patriotiques sont des symboles importants. Nous y sommes tous attachés ; nous sommes tous des défenseurs actifs de la mémoire de toutes les générations du feu. cet attachement qui nous réunit aujourd'hui. C'est l'estime et l'admiration que nous portons au monde combattant, aux femmes et aux hommes qui ont servi et qui servent notre pays, qui nous rassemblent. Mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs, je vous remercie du fond du coeur de votre intérêt pour les questions liées au monde combattant et à ses associations. Je loue votre souci de préservation de la mémoire et de mise en valeur des drapeaux associatifs. Ces femmes et ces hommes, nous les rencontrons dans nos territoires, nous participons à leurs réunions, nous partageons avec eux des moments d'unité lors des commémorations et des journées nationales. Les porte-drapeaux y occupent une place singulière. Au sens propre, ils portent la Nation. Je les en remercie chaque fois que je les rencontre. Ils sont de toutes les générations. En novembre dernier, dans les Ardennes, lors des commémorations du centenaire de l'armistice de 1918, j'ai rencontré un jeune écolier qui tenait son rang parmi les porte-drapeaux.

que je voulais mettre en valeur, car je crois qu'il faut être optimiste et convaincu que la transmission et la perpétuation de la mémoire combattante sont déjà sur de bons rails.

Ainsi, la disparition des deuxième et troisième générations du feu d'ici à quelques années aura pour conséquence la disparition d'associations d'anciens combattants. Nous nous y préparons. Cette proposition

de nombreuses problématiques abordées étant d'ores et déjà traitées par des textes et des règlements en vigueur. Souvent, le droit comme la pratique actuelle permettent de répondre à ces situations.

en l'absence de précision sur la dévolution des biens dans les statuts de l'association, l'assemblée générale décidant la dissolution doit statuer sur ce point. Si tel n'est pas le cas, le décret du 16 août 1901 pris pour l'exécution de la loi du 1 juillet 1901 prévoit la nomination d'un curateur chargé de convoquer ladite assemblée générale.

Aujourd'hui, si un drapeau, propriété d'une association, est trouvé entre les mains d'une autre personne, la loi dispose que l'association peut légitimement revendiquer le drapeau dans un délai de trois ans.

qui ne semble justifié par aucun motif d'intérêt général. La frontière est mince avec la privation pure et simple du droit de propriété sans indemnité,

nous ont confirmé qu'ils ne souhaitaient pas ce dispositif, le jugeant inutile et contraignant. En effet, certaines associations ont déjà mis en place des dispositifs internes, qu'elles estiment efficaces et suffisants.

le groupe de travail que j'évoquais à l'instant est complètement mobilisé sur cette question. Nous y travaillons en parfaite concertation avec les associations, à leur demande d'ailleurs, car elles sont bien conscientes que leur avenir pourrait être difficile.

faut-il rappeler ici, au Sénat, combien les associations d'anciens combattants sont un vecteur essentiel de la transmission de la mémoire collective ? Nous sommes nombreux à les côtoyer régulièrement sur le terrain, en tant qu'élus locaux. Nous connaissons la qualité et la vitalité de leur engagement pour relayer cette mémoire combattante qui nous est si chère. Que ce soit lors des commémorations qui jalonnent le calendrier national ou lors de leurs assemblées générales, les associations d'anciens combattants honorent toujours, par leur présence encore active, nombre de villages et de villes de France. Le jour viendra où le dernier combattant de la Seconde Guerre mondiale, puis celui de la troisième génération du feu, s'éteindront. Le dernier Poilu nous a quittés en 2008. Selon la dernière prospective sur l'évolution du nombre de ressortissants de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, les anciens combattants auront perdu plus du tiers de leur effectif entre 2013 et 2023. Dans ces conditions, on le sait, nous assistons à l'extinction progressive de la majorité des associations d'anciens combattants qui s'étaient constituées au lendemain de la Première Guerre mondiale.

la dissolution ou la fusion d'une association affectant parfois le sort des étendards jusqu'alors arborés fièrement par les porte-drapeaux qui avaient le privilège d'exercer cette fonction honorifique. La dimension symbolique des drapeaux d'associations d'anciens combattants, que chacun d'entre nous mesure bien, mérite une attention toute particulière. À cet égard, je salue l'initiative de notre collègue Françoise Férat, qui s'est faite, si j'ose dire, la porte-voix de cette cause qui fait consensus. En effet, il est choquant de retrouver les drapeaux d'associations d'anciens combattants sur les étals des brocantes et des vide-greniers ou sur les sites de vente en ligne. Si l'on peut comprendre l'intérêt d'un public passionné

La charge historique et émotionnelle que véhiculent ces drapeaux impose d'assurer une protection que le droit actuel ne permet pas suffisamment. L'auteur de la proposition de loi l'a très justement rappelé. Le texte initial prévoyait un dispositif unique pour, d'une part, organiser la restitution des drapeaux d'associations d'anciens combattants, et, d'autre part, en interdire la vente. La commission, sous l'impulsion pertinente de Mme la rapporteure, l'a récrit afin de contourner les difficultés liées au droit de propriété garanti par la Constitution, en proposant notamment une exception à la prescription acquisitive pour les drapeaux portant les signes distinctifs d'une association. Madame la rapporteure, le RDSE approuve, bien entendu, le texte issu des travaux de la commission, qui respecte l'intention initiale des auteurs de la proposition de loi, à savoir la protection des drapeaux, ainsi que leur restitution aux associations, aux communes ou aux écoles. Pour ma part, je proposerai un amendement, soutenu par mon groupe, visant à mentionner clairement les musées comme des destinataires éventuels de ces drapeaux. Ils sauront eux aussi les valoriser au profit de la mémoire nationale.

et toutes proportions gardées, j'ajouterai qu'il faut continuer de sortir les drapeaux, car ils ne sont pas seulement le témoignage d'un passé révolu ; ils sont aussi le rappel des valeurs de fraternité et de solidarité dont nos sociétés ont toujours grandement besoin. Dans un contexte où le service militaire n'existe plus, où le rapport au temps a changé pour plus d'immédiateté, où d'autres mémoires, tout aussi légitimes, émergent, il n'est pas facile de perpétuer la mémoire combattante auprès des jeunes. Si elle est éternellement gravée dans le marbre des monuments aux morts ou des mémoriaux, il faut aussi s'employer à la rendre vivante, pour que les anciens combattants ne soient pas uniquement un souvenir d'hier, mais aussi le symbole de notre liberté d'aujourd'hui. Il est par conséquent important de soutenir toutes les démarches qui apportent une pierre supplémentaire à la politique de mémoire que mènent au quotidien l'État, les collectivités locales et leurs élus, ainsi que les associations.

cette proposition de loi qui contribue à l'entretien de la mémoire combattante et qui instaure le respect de tous les drapeaux qui la représentent. La

Ils étaient vingt et trois quand les fusils fleurirent « Vingt et trois qui donnaient leur coeur avant le temps « Vingt et trois étrangers et nos frères

chers collègues, ces vers de Louis Aragon célèbrent la mémoire des résistants du groupe Manouchian, principale force d'opposition directe aux Allemands en région parisienne, des partisans dotés d'un courage sans faille, qui furent fusillés le 21 février 1944 au Mont-Valérien. Alors que le dernier de ses membres s'est éteint en 2018, le devoir de mémoire, les 35 000 monuments aux morts et ces quelques vers restent les derniers remparts contre l'oubli des « grands anciens », ces morts pour la patrie qui ont sacrifié leur vie pour rendre la nôtre possible. La proposition de loi que nous examinons aujourd'hui vise à protéger les drapeaux des associations d'anciens combattants en créant une présomption de propriété au profit de ces Elle prévoit également le transfert des drapeaux, en cas de dissolution de l'association ou sur décision de son assemblée générale, à la commune compétente, chargée de relayer, auprès d'associations actives ou d'établissements scolaires, le devoir de mémoire des anciens combattants. Enfin, une association d'anciens combattants, une fédération ou la commune pourra obtenir gratuitement la restitution d'un drapeau détenu par un particulier. Nous soutenons pleinement cette initiative et saluons le travail de la sénatrice Françoise Férat. Le réseau d'associations dont il est question s'est structuré dès l'année 1915 pour faire reconnaître les droits matériels et moraux des anciens combattants, des mutilés, des « gueules cassées », des démobilisés de la Grande Guerre. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, plus de 10 000 associations d'anciens combattants étaient actives sur le sol national. Chacune d'entre elles possède ses propres symboles, son drapeau tricolore chargé d'histoire et brodé de lettres d'or. Elles regroupent les anciens combattants des deux guerres mondiales, des guerres du Golfe, d'Algérie, de Yougoslavie, d'Afghanistan, et contribuent au devoir de mémoire reliant passé et présent. Permettre à des générations de Français de mieux comprendre l'histoire de la France, d'en mesurer les sacrifices, de s'imprégner des valeurs républicaines pour éclairer leur avenir, leurs choix, leurs engagements tels sont les enjeux du devoir de mémoire, que Simone Veil proposait de remplacer par un devoir d'histoire, articulant souvenir et transmission. « La patrie ne s'apprend pas par coeur, elle s'apprend par le coeur », disait Lavisse. Elle s'apprend par la résonance à travers les siècles de ces noms d'hommes et de femmes qui se sont engagés pour défendre la vie, la liberté, l'avenir de la France. Ces noms, trop souvent, tombent dans l'oubli. Qui se souvient de Jeannette Guyot ? À 20 ans, elle traversait les bois et les champs dans la nuit silencieuse, suivie d'enfants, d'hommes et de femmes, les emmenant loin de la terreur. Jeannette Guyot, parachutée en bord de Loire pour repérer les zones de largage en vue du débarquement. Jeannette Guyot, ouvrant une antenne de radio clandestine à Paris, dans un tabac, à deux pas d'un bureau de la Gestapo ... Seul un article d'un journal britannique annonça sa mort, le 10 avril 2016 ! En France, il n'y eut pas un mot dans la presse, à la radio, sur les réseaux pour lui rendre hommage. Comprendre le passé, le regarder avec lucidité pour en saluer les grandes heures, sans renier les heures sombres, ce sont les conditions indispensables pour bâtir sur l'exemple. En honorant la mémoire des héros de la Nation, la commémoration anime un lien qui libère, érige un signe de concorde entre les générations Il est bien sûr du devoir de l'État, de la puissance publique en général, de maintenir cette mémoire vive, à l'image de la flamme du souvenir toujours entretenu, veillant nuit et jour la tombe du Soldat inconnu, sous l'Arc de Triomphe. À l'heure où les symboles de la mère patrie sont tagués, dévastés, pris d'assaut par des casseurs bêlants, où le poison rampant de l'extrémisme se répand à travers une Europe fragilisée, où le communautarisme divise la France en son coeur, il nous faut veiller à maintenir vivants les souvenirs de notre histoire commune, à replacer les symboles de la République au centre de nos villes, de nos villages, dans nos écoles et nos mairies. Chers collègues, les drapeaux des associations d'anciens combattants sont de ces symboles que nous avons la responsabilité de protéger. Il y va à la fois de notre héritage

Nos condoléances vont également à ses frères d'armes qui poursuivent un difficile combat contre le terrorisme islamiste dans la bande sahélo-saharienne. De même, je tiens à rendre hommage aux associations d'anciens combattants, tant pour leur travail patient auprès de ceux qui ont payé un lourd tribut à la Nation que pour leur contribution au devoir d'histoire et de mémoire. C'est une évidence, ces associations participent à la transmission de la mémoire et des valeurs de notre pays. À l'échelle de nos territoires, elles oeuvrent en faveur d'un maillage de la perpétuation du souvenir. Je veux remercier à mon tour François Férat et Élisabeth Doineau pour leurs travaux et leur capacité d'écoute. Beaucoup d'entre nous ont été sollicités à propos des difficultés relatives à la protection des drapeaux d'associations d'anciens combattants.

Emblèmes de la Nation française, ils témoignent de l'engagement patriotique des territoires composant la France qui ont participé aux épreuves de la guerre et à la défense de notre pays. Cependant, beaucoup d'associations d'anciens combattants sont dissoutes du fait de la disparition de leurs membres, qui, ne l'oublions pas, étaient autant de délégués précieux et directs de cette mémoire dont la transmission doit Rien ni personne n'échappant aux outrages du temps qui emporte tout, y compris ce que les hommes peuvent avoir de plus précieux, il n'est pas surprenant que des drapeaux puissent être proposés à la vente. Cela peut apparaître comme une double offense : offense à la mémoire de ceux qui les ont portés, offense à la mémoire des anciens combattants qu'ils représentent. Pour autant, leur vente n'est nullement illégale. Plus largement, il nous faut répondre à la question du devenir des objets mémoriels et de leur marchandisation éventuelle, qui peut parfois poser d'importants problèmes éthiques. Pour le cas particulier des drapeaux d'associations d'anciens combattants, il revient au législateur d'organiser leur conservation dans une logique de préservation et de transmission de la mémoire, sans pour autant entraver le droit de propriété et possession, ainsi que la prescription acquisitive. Je salue donc l'initiative de notre collègue Françoise Férat, qui nous a permis d'aborder cette question. Toutefois, interdire à son propriétaire légitime de vendre un drapeau ayant appartenu à une association d'anciens combattants serait de nature à mettre en cause le droit de propriété, droit fondamental inscrit dans notre Constitution. De fait, nous sommes satisfaits de la solution juridique proposée par notre rapporteure. La création d'une exception au principe de la prescription acquisitive pour les associations leur permettra, d'une part, de conserver la propriété des drapeaux grâce à la présomption de propriété, et, d'autre part, de se les faire restituer gratuitement, ce qui est important, car leurs moyens sont limités. Enfin, je salue l'alinéa relatif à la « conservation » des drapeaux en cas de dissolution des associations. Leur transmission à la commune de domiciliation permettra au territoire de conserver ce qui n'est autre qu'un témoignage de sa propre histoire. Quant à la possibilité de les confier à un établissement scolaire ou à une association, c'est également une très bonne chose, un moyen de donner une deuxième vie à ces drapeaux et, ainsi, de prolonger l'oeuvre de mémoire auprès des générations suivantes.

On en retient généralement que « la Nation est une âme, un principe spirituel » et qu'elle se perpétue par « le consentement actuel, le désir de vivre ensemble, le plébiscite de tous les jours », mais on oublie trop souvent que Renan ajoutait que si cette âme, si cette âme, ce principe spirituel trouve sa force et sa légitimité dans le présent, il le trouve aussi dans le passé, ce passé qu'il qualifiait de « possession en commun d'un riche legs de souvenirs » alimenté alimenté par « la volonté de continuer à faire valoir l'héritage qu'on a reçu indivis [ ...] lui-même constitué par le sentiment des sacrifices qu'on a faits et de ceux qu'on est disposé à faire encore. » De ce point de vue,

Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, madame la rapporteure, mes chers collègues, la proposition de loi de notre collègue Françoise Férat vise à protéger le devenir des drapeaux des associations d'anciens combattants en interdisant leur vente. Dans cette perspective, le texte adopté par la commission prévoit le transfert à la commune des drapeaux appartenant à une association d'anciens combattants

Dans le cas où un porte-drapeau décède, les drapeaux qu'il conservait devront être restitués aux associations d'anciens combattants, à leurs « ayants droit » ou à toute personne attachée au devoir de mémoire et au souvenir. L'alinéa 5 de l'article unique crée judicieusement, me semble-t-il, une présomption de propriété pour les drapeaux portant les signes distinctifs d'une association d'anciens combattants. d'une association d'anciens combattants. L'alinéa suivant permet à une association d'anciens combattants ou, à défaut, à une fédération ou à la commune dans laquelle l'association était domiciliée d'obtenir gratuitement qu'un drapeau se trouvant entre les mains d'un particulier lui soit restitué. Il s'agit à la fois de prévoir les règles applicables en cas de disparition de la personne ou de l'association conservant des drapeaux et de prévoir des sanctions pour garantir leur application. Ce texte couvre l'ensemble des hypothèses possibles afin de protéger cette part incontournable de notre patrimoine mémoriel. Sur le plan des sanctions, le texte initial

punie de trois ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende. Autrement dit, le droit existant comporte déjà une mesure coercitive garantissant au mieux l'application des dispositions de ce texte. De plus, nous sommes toutes et tous ici d'accord pour reconnaître que ces drapeaux constituent un symbole fort de l'histoire de notre pays. Aussi cette partie de notre héritage est-elle à préserver et à transmettre. C'est pourquoi je tiens à insister sur le bon sens dont témoigne cette proposition de loi qui « laisse ouverte » la possibilité de léguer ces drapeaux à d'autres associations d'anciens combattants ou à des établissements scolaires et qui encourage les communes à le faire. Au-delà de la question du devenir des drapeaux, cette proposition de loi prend en compte la problématique de la protection de notre histoire et vise à adapter notre politique mémorielle, qui s'appuie largement sur les associations d'anciens combattants,

À ce titre, les ventes de drapeaux d'associations d'anciens combattants dans les brocantes ou sur internet mettent en péril notre patrimoine mémoriel. Il est donc indispensable d'en finir avec cette marchandisation et cette liquidation des emblèmes des conflits passés.

En effet, le patrimoine mémoriel peut être considéré comme faisant partie du patrimoine culturel. Les modifications du texte proposées par la commission permettront de limiter, malgré tout, les ventes de drapeaux d'associations d'anciens combattants, en prévoyant au bénéfice acquisitive. Ainsi, si un particulier possède un drapeau d'une association d'anciens combattants, il pourra lui être demandé à tout moment de le remettre à cette association. Désormais, dès lors qu'un drapeau portera les signes distinctifs d'une association d'anciens combattants, il sera présumé appartenir à cette association, sauf preuve du contraire. Les associations pourront récupérer gratuitement leurs drapeaux qui viendraient à être vendus indûment. C'est une mesure de sécurité indispensable dès lors que la vente des drapeaux demeure autorisée. Afin de garantir la préservation de notre patrimoine, les drapeaux d'associations dissoutes pourront être transférés à la commune de domiciliation. La proposition de loi relative à la protection des drapeaux des associations d'anciens combattants va donc renforcer la sauvegarde de notre mémoire. de l'examen de ce texte pour rappeler au Gouvernement, qui a diminué les crédits alloués à la politique de mémoire de 2,79 millions d'euros en 2019, soit de plus de 20 % par rapport à 2018, que la protection de notre mémoire passe également par l'arrêt des réductions de budgets. Si l'on souhaite prévenir la marchandisation des drapeaux sur les marchés, il faut aussi maintenir les subventions aux associations d'anciens combattants ! Je pense, en particulier, à l'Association républicaine des anciens combattants, l'ARAC, dont l'État a supprimé la subvention d'action sociale de 70 000 euros.

En conclusion, pour l'ensemble des raisons que je viens d'évoquer, le groupe communiste républicain citoyen et écologiste votera en faveur de

je suis née dans un territoire, le Calvados, riche d'histoire, de moments glorieux et d'autres plus douloureux. Dans mon département, que je représente ici, le rôle des associations d'anciens combattants n'est plus à démontrer, tant il est essentiel. Elles assurent régulièrement les commémorations patriotiques qui rythment la vie de nos communes, de nos villages, et font un travail remarquable auprès des plus jeunes générations, rappelant sans cesse que la liberté dont elles jouissent aujourd'hui est due au sacrifice de beaucoup de leurs aînés. Tout doit être entrepris pour faire vivre la mémoire combattante. Malheureusement, nos anciens combattants des deuxième et troisième générations du feu s'éteignent progressivement. De fait, les associations représentatives du monde combattant ont tendance à disparaître et, avec elles, leurs drapeaux. Oubliés au fond d'un grenier, parfois vendus par les familles d'anciens combattants, ces drapeaux doivent être mieux protégés, afin que le souvenir qu'ils entretiennent ne s'efface jamais. Rappelons Rappelons d'ailleurs qu'un porte-drapeau n'est pas le propriétaire du drapeau et qu'il n'a donc pas à décider de l'avenir de cet emblème, et ses proches encore moins. La proposition de loi qui nous est aujourd'hui soumise est le fruit du large consensus dont le Sénat sait faire preuve sur la question de la mémoire combattante. Elle vise

à la dimension patriotique et symbolique forte ! Je me rappelle très bien, par exemple, l'émotion qui a été la mienne, en juillet 2015, lorsque le drapeau hissé à la libération de Caen, en 1944, s'est mis à flotter de nouveau au vent lors de la cérémonie commémorative. Il avait disparu depuis soixante et onze ans ... La version initiale de la proposition de loi de Mme la sénatrice Françoise Férat posait un certain nombre de difficultés juridiques, notamment parce qu'elle portait atteinte aux droits attachés à la propriété. Il convenait d'y remédier. Dans sa version issue des travaux de la commission des affaires sociales, le texte prévoit désormais le transfert à la commune des drapeaux appartenant à une association d'anciens combattants, en cas de dissolution de celle-ci et à défaut de dispositions statutaires ou de décision de l'assemblée générale Il crée par ailleurs une présomption de propriété lorsqu'un drapeau porte les signes distinctifs d'une association d'anciens combattants. Il permet également à cette dernière, ou sinon à une fédération ou à la commune dans laquelle l'association était domiciliée, d'obtenir qu'un drapeau se trouvant entre les mains d'un particulier lui soit restitué alinéa de l'article unique de la proposition de loi rappelle la possibilité, pour une commune qui serait devenue propriétaire d'un drapeau d'association d'anciens combattants, de le confier, par exemple, à un établissement scolaire ou à une autre association représentative du monde combattant, afin d'en assurer la conservation. Tout cela va dans le bon sens pour la politique mémorielle de la France, sans contrevenir au principe d'indépendance du monde associatif. Je ne peux terminer mon intervention sans remercier les représentants calvadosiens

Si l'organisation d'une cérémonie internationale en présence notamment de chefs d'État semblait une évidence, c'est plutôt l'incertitude et l'incompréhension qui dominent aujourd'hui localement, le lieu de cette cérémonie n'étant toujours pas connu situation est mal vécue par les associations représentatives du monde combattant, par les élus et, plus largement, par la population calvadosienne dans son ensemble, très attachée à ces cérémonies. Il devient urgent qu'une décision soit prise, afin que les différentes parties prenantes puissent s'organiser, et ainsi rendre compte de l'importance de ce qui s'est passé, sur nos plages, pour libérer l'Europe occupée, le 6 juin 1944, et rendre hommage à ceux qui ont combattu et, pour beaucoup, sacrifié leur vie.

C'est donc bien un symbole qui est en jeu, pour notre pays mais également pour nos communes. Ne l'oublions pas, les drapeaux des associations du monde combattant constituent un héritage. Il convient de les préserver.

engagés sur le front pour repousser l'ennemi et pour que la bannière de notre pays continue de flotter. Beaucoup ont même donné leur vie pour la liberté, pour la fraternité de notre peuple. À travers ces cérémonies, locales et nationales, nous mettons en avant leur engagement, mais aussi celui de ces femmes faisant vivre leur famille et jouant un rôle indispensable dans les campagnes, les hôpitaux, sans oublier l'économie du pays. C'est bien leur courage qui rayonne à travers ces drapeaux ! Mais, permettez-moi de le souligner, en cette période de conflits et de tensions, le texte soumis à nos débats revêt une tout autre dimension. Certains, il faut le dire, le dire, s'en prennent sans vergogne aux symboles de la République, à nos forces de l'ordre, d'autres brûlent des véhicules de la force Sentinelle ou dégradent des lieux historiques. Je pense notamment à l'Arc de Triomphe, qui, érigé au lendemain de la bataille d'Austerlitz,

! En ces temps troublés, il est urgent de revenir aux fondamentaux et de rappeler l'importance de ce travail de mémoire pour nos combattants d'hier et d'aujourd'hui. Oui, c'est bien l'esprit du souvenir qui doit ranimer notre société, ce même esprit qui a fait naître ces associations que nous défendons par le biais de ce texte. Leur vocation était de passer le témoin aux générations suivantes et de rappeler que la liberté se gagne au prix le plus fort.

Je le disais à l'instant, c'est une émotion, mais aussi une fierté. Ce drapeau a perduré malgré les épreuves et il continuera à flotter en dépit des vents et des tempêtes de l'histoire. Cependant, il est regrettable de devoir constater la disparition d'objets liés à ces associations, comme le rappelait notre collègue rapporteure Élisabeth Doineau. Moralement, cela suscite une inquiétude. Mes chers collègues, il nous faut être attentifs à cette situation : un drapeau, ce n'est pas n'importe quel symbole, ce n'est pas n'importe quel bien ; c'est l'âme d'une nation, ce sont les couleurs d'un peuple, c'est le témoin de notre histoire commune. En se battant pour la patrie, des hommes l'ont brandi avec fierté. Par conséquent, nous devions nous pencher sur les cas de revente de drapeaux d'associations d'anciens Il nous appartient, en tant que législateur, d'y veiller. Tel est l'objectif atteint au travers de cette proposition de loi. Ainsi, grâce à l'adoption de ce texte, le drapeau qui portera les signes distinctifs d'une association d'anciens combattants sera présumé lui appartenir. Par ailleurs, l'association originellement propriétaire d'un drapeau vendu dans une foire, sur un marché ou à l'occasion d'une vente publique, voire sur internet, la fédération d'associations à laquelle elle appartenait ou, à défaut, la commune dans laquelle elle était domiciliée, pourra se le faire rendre à titre gratuit. Ce sont des dispositions importantes, qui visent à protéger les associations et à les valoriser dans leur action. En outre, ce texte n'oublie pas les communes. Ainsi, en cas de dissolution d'une telle association, à défaut de dispositions statutaires ou de décision de l'assemblée générale, ses biens seront transférés gratuitement à la commune de domiciliation. Celle-ci pourra d'ailleurs confier les drapeaux à un établissement scolaire ou à une autre association d'anciens combattants,